La séance est reprise, nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'amendement 357 article additionnel après l'article 11 qui est-ce. Donc cet amendement 357 et présenté par Madame de Marco, qui a la parole. Merci, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, pour encourager le développement des énergies renouvelables, y compris sur les bâtiments situés dans des espaces protégés, voici un amendement qui vous propose que je vous propose d'adopter, qui vise à rendre obligatoire la réalisation d'une étude de faisabilité sur le potentiel d'énergie renouvelables lorsqu'un espace protégé subi une opération de restauration de réparation ou de modifications. Qu'est l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci président écoutez je peux reprendre les commentaires que j'ai fait avant la pause, c'est un avis défavorable sur cet amendement. Le ministre, c'est un avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Donc Donc il est pas adopté. Je me voir article 11 sexy nouveau qui est pour.

Monsieur Lahellec d'accord et il y a un amendement identique présentée par le gouvernement, Madame la Ministre, le six Cet amendement propose la suppression de l'article onze ces pièces qui prévoit des avantages fiscaux pour les entreprises qui installent des systèmes de production de production d'énergie renouvelable sur toiture la production d'énergie renouvelable en toiture, via des panneaux football. Daïc ou solaire thermique et déjà aidé par des tarifs spécifiques comme les tarifs d'achat pour l'électricité, par ailleurs, l'article onze ces pièces prévoit également que le dispositif des certificats d'économie d'énergie puisse financer l'installation de dispositifs de production d'électricité renouvelable en remplacement d'une production électrique non renouvelable, les ses 2 E régis par la législation européenne et nationale certifie des économies d'énergie, et non des substitutions énergétiques cela et donc incompatible avec la législation européenne et nationale des dispositifs de financement adaptés existent déjà pour ces installations, c'est pourquoi je vous invite à adopter cette avant qui permet d'avoir des modes de financement qui sont réguliers et compatible avec le droit. Oui, je lui ai donné un avis défavorable à à ces deux amendements, nous avons remporté renforcer les obligations de couverture de existant existants et de nouveaux donc il nous paraît important, en contrepartie d'accompagner ceux qui investissent et même si, effectivement, des aides existent déjà : le suramortissement est une opération intéressante pour accélérer le développement des énergies renouvelables et puis quant au CE, les règlements sont faits pour évoluer, donc j'ai, j'espère qu'avec ce que nous avons intégré dans le texte, ce sera le cas dans, dans, dans un temps relativement proche donc c'est un avis défavorable. Je mais au voir cet amendement, sauf il y a pas de demande d'explications de vote dans quels sont ceux qui sont favorables à ces amendements de suppression.

Quels sont ceux qui sont contre. Ils sont adoptés. Du coup, il y a pas de vote sur l'article qui est supprimé. Après le onze, ces pièces, nous avons à l'amendement numéro 280 présenté par Monsieur Gontard.

ce tarif doit pouvoir s'appliquer de façon identique à toutes les opérations d'autocollants consommation qui sont définies dans le code de l'énergie, et cela, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, donc c'est un amendement qui est proposée par l'association s qui vise donc à développer cette auto-consommation. Monsieur rapporteur favorable à l'eau de consommation et tout ce qui peut quand même de la développer, donc c'est un avis favorable à cet amendement. Madame la ministre est l'avis du gouvernement. C'est un avis défavorable, les auto-consommateurs individuels sont actuellement exonérés d'assises sur l'électricité sur la part qu'ils auto-consomme car cette électricité ne transite pas sur le réseau public de distribution d'électricité, cela n'est naturellement pas le cas de l'électricité autant consommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, c'est pourquoi une telle exonération ne sauraient être mises en oeuvre, hé oui, le l'électricité transite bien par le réseau et donc doit pas en prendre sa part dans la rémunération du réseau. Je soumets au Sénat, l'amendement 280 quels sont ceux qui sont pour.

un amendement portant article additionnel de Madame Préville le 77, madame, vous avez la parole. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le seuil de 3 kilowatts crête, a été mis en place en 2008 à une époque où la recette annuelle générées par une installation de cette puissance était de l'ordre de 1800 euros pour un ensoleillement correspondant à la moyenne nationale, or compte tenu de la baisse des tarifs d'obligation d'achat enregistrée depuis cette époque, une installation équivalent génère en 2022 une recette de seulement 600 euros porter le plafond d'exonération pour les seules installations mises en service à partir du premier je vais 2023 à 9 ce que je propose dans cet amendement, qui correspond à un seuil figurant dans les arrêtés tarifaires est de nature à augmenter sensiblement, mais à coût maîtrisé la quantité d'électricité produite par les particuliers tout en optimisant à la fois les surfaces mobilisables en toitures des maisons individuelles et les capacités d'accueil du réseau public de distribution sans travaux de renforcement. C'est un avis défavorable puisque, s'agissant des installations de 3 à 9 kWc étant donné leur surface correspondant souvent les personnes qui en bénéficient correspondent souvent à des entreprises, la cibles serait donc différente que celle visée autrement et votre amendement conduirait de facto quasiment à supprimer l'exonération actuel car il ne pourrait s'appliquer qu'aux revenus générés par l'électricité vendue dans le cadre d'une opération d'autoconsommation qui est limitée, comme vous venez de le souligner il complexe et retiré beaucoup la situation existante pour de nombreux petits producteurs, j'ajoute que sur l'autoconsommation des décisions récentes ont été prises pour faciliter le financement de ces dispositifs donc je veux le signaler, elles ont été passés au Conseil supérieur de l'énergie ont donné lieu à des à des textes réglementaires qui permettent notamment de préfinancer, les investissements d'autoconsommation là où vous savez c'était divisé sur 5 années, là on verse 80 dès la première année de l'investissement et ils nous avons également favoriser l'autoconsommation collective qui était effectivement le parent pauvre de l'autoconsommation, il y a bien une action en faveur de l'autoconsommation, et je pense qu'elle permet de répondre aux objectifs que vous poursuivez, ce sont des textes qui datent de septembre ou d'octobre je regarde mes équipes, hein, c'est ça : septembre. Monsieur Salmon. Salmon. C'est une incompréhension. Donc je soumets à l'Assemblée, l'amendement 377 pardon qui a fait l'objet d'avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour.

Merci monsieur le Président, répondre à au au projet de photovoltaïque qui sont peut être d'envergure, un peu moins large que ce qu'on a pu traiter jusqu'alors donc, si le potentiel est en effet très important de ces projets, il semble utile aussi de traiter également les enjeux relatifs à l'autoconsommation la PPE, considère que l'autoconsommation est une pratique destiné à se développer et à prendre une place de plus en plus prégnante dans le mix énergétique dans les années à venir, c'est en effet une pratique qui peut permettre aux ménages les plus modestes de devenir acteurs de leur propre qu'on se production et consommation d'énergie tout en réduisant leurs dépenses en la matière, pour autant, les aides existantes pour accompagner l'installation de panneaux photovoltaïques en vue d'une opération d'autoconsommation sont complexes à mobiliser et ne couvre pas la totalité des investissements nécessaires, l'éco-prêt à taux zéro mis à la disposition des particuliers qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique permet d'obtenir après allant de 7 à 30000 euros aussi, cet amendement vise à ouvrir l'éco-PTZ aux travaux d'installation de panneaux solaires permettant l'autoconsommation, c'est l'objet de cet amendement, je vous remercie.

c'est une demande de retrait sinon rejet puisque comme je voulais, a indiqué : nous avons d'autres mesures qui permettent de soutenir. L'autoconsommation un arrêté tarifaire fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par des installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance inférieur à 500 il prévoit une prime à l'investissement, un appel d'offres pour les installations photovoltaïque en autoconsommation supérieur toute aide supplémentaire devrait conduire à une déduction d'autant sur les dispositifs susmentionnés, comme vous le savez l'effet global serait donc neutre pour le client, tout en ajoutant une complexité administrative enfin je redis les dispositifs que nous venons de prendre pour favoriser l'autoconsommation et l'autoconsommation collective. Monsieur Dantec demande, a expliqué son vote. Oui merci monsieur le président moi je, je soutiendrai l'amendement de Madame Loisier, l'explication qui vient de nous être donné, je pense que derrière il y a un point absolument stratégique et que vous avez souligné madame la ministre. On est là pour économiser l'argent de l'État. Dans un certain nombre de domaines, on a plus besoin de subventions, on a besoin d'accès à des prêts qui se remboursent pas le tarif d'achat simplement c'est sur l'accès au prêt qu'on a énormément difficultés y compris toutes les classes moyennes qui veulent mettre du panneau photovoltaïque qui vont voir leur banque et qui ont acheté une maison sont déjà au 30 35 % de taux d'endettement et n'ont pas accès auprès alors qu'il y a un modèle économique derrière et qui a absolument pas besoin de subventions et de la subvention pour des ménages qui ont peu de liquidités, ça ne marche pas, donc derrière l'amendement qui est là, c'est un vrai changement de stratégie c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de subventions, on a besoin d'accès à des prêts qui se rembourse sur des modèles économiques robustes aujourd'hui les co-PTZ est au coeur de ça, donc il nous faut effectivement faciliter l'accès auprès et ça fera des économies de subventions pour l'État. Madame Bio. Juste dire que j'ai entendu les explications de Madame la Ministre, mais je remercie le le rapporteur pour cet avis positif cet amendement, il a pour objectif de de faire que les énergies renouvelables, elle soit accessible pour tous, toutes les bourses, en réalité, donc je comprends vraiment pas l'avis défavorable et je je remercie la commission et le rapporteur pour cet avis favorable merci. Donc, nous votons sur l'amendement 186 qui qui est maintenu avec un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté sur l'article 11 pièces, nous avons un amendement de suppression du gouvernement qui, le 598. Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 oct Yes par là. Commission car celui-ci exclut la possibilité laissée aux pouvoirs réglementaires de déterminer si le bénéfice de l'article L 116 et limiter ou non à l'auto-consommation si une réflexion doit pouvoir être engagée sur cette limitation, il convient d'expertiser l'encadré afin d'éviter le développement de construction Libye dont le seul objet serait en réalité la production d'énergie limite considérablement la capacité des collectivités d'encadrer la délivrance des autorisations d'urbanisme pour un projet comportant un dispositif de production d'énergie renouvelable en imposant que ces prescriptions ne conduise pas à un renchérissement du coût du projet hors des prescriptions notamment parfaitement justifiée pour garantir la bonne intégration architecturale ou paysagère. On en a suffisamment parlé des secteurs sensibles du Patrimoine de de la bonne intégration dans des villages de caractère ou le plus souvent un surcoût, même lorsqu'il est modéré, un tel mécanisme sous prétexte de faciliter le développement des ENR sur les constructions et donc susceptible d'aboutir exactement à l'effet inverse et ça diminuerait diminuerait l'acceptabilité des projets comportant des ENR, pour cette raison fondamentale, je propose la suppression de l'article 11 oct hôtesse. L'avis de la commission sur portable. C'est un un avis évidemment défavorable à cette demande de suppression de l'article 11 oct y a ceux qui intègrent un certain nombre de d'éléments sur lesquels je vais, je vais pas revenir, mais ce serait voilà, remettre en cause ce qui a été convenu c'est donc un avis défavorable. Je mets aux voix un amendement de suppression 598 faisant l'objet d'un avis défavorable de la commission, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre n'est pas adopté ensuite 2 amendements font l'objet d'une discussion commune d'abord le 416 madame Préville. Merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 11 obtiennent instaure l'obligation pour les nouveaux bâtiments d'être conçue pour être en mesure d'accueillir un système de production d'énergie renouvelable, ce qui est une excellente chose, cette mesure constitue en effet une avancée importante, mais pour s'assurer qu'elle soit réellement opérationnel, il convient de préciser, d'une part que l'intégration proprement dit, d'un tel système peut être immédiate ou future, c'est-à-dire la notion de bâtiment sous Larisa Blue Solar Eddy, d'autre part que le réseau électrique intérieure du bâtiment doit être conçu et dimensionné en conséquence, que ce soit au niveau du tableau électrique pour une maison individuelle ou du dernier étage d'une colonne montante dans le cas d'un immeuble collectif à plusieurs étages. Et en discussion commune là cet amendement 271 de Monsieur Gontard qui est défendu. Par lui même. Merci monsieur le le président. Cet amendement vient préciser, en fait, l'excellente disposition de de cet article qui a été ajouté en commission, en indiquant que les caractéristiques Nick techniques garantissant l'intégration de de procédés de production d'énergie rouvre Venables doit figurer au au permis de construire, en effet, on trouve plutôt intéressant d'avoir cette obligation technique de faire en sorte que notamment des panneaux solaires, soit intégrés pour toute forme de de construction et mais ça nous semblait intéressant que ça puisse être intégrée dans les dans les permis de construire, ce qui permettait

C'est un avis défavorable pour les raisons que j'ai exprimé étant défavorable, déjà à l'article je suis défavorable aux amendements complémentaires. Donc, nous commençons par l'amendement 416 et retiré il retiré d'accord.

madame, monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement a pour but de préciser effectivement que d'évaluer les conditions à la fois économiques mais aussi les conditions physiques ne supporte habilité des toitures dans le cadre de du changement des toitures amiantés par une production énergétique à partir de photovoltaïque. L'avis de la commission. Oui c'est un avis favorable parce que c'est une précision importante : il y a un potentiel sur les toits de plusieurs centaines de milliers et effectivement, avant d'aller chercher des surfaces autre concentrons-nous donc ce rapport est important pour permettent de déterminer ce ce ce désamiantage des, des, des toitures au travers de voilà de cette étude approfondie. Oui, le gouvernement, c'est un avis défavorable, puisque nous étions défavorables sur l'article 11 nièce. L'amendement 486 avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Contre. Il est adopté ensuite l'amendement 273 du président Gontard, merci Monsieur le Président, des toitures amiantés et je pense que dans cette, dans cette perspective, il nous semblait intéressant que soit précisée justement dans les éléments qui seront, qui seront réfléchis et qui seront analysés dans ce rapport que il y a un recensement par la puissance publique de des toitures amianté de plus de plus de 150 mètres carrés, on voit bien qu'on a une vraie problématique sur l'ensemble de ces toitures souvent agricoles, mais pas que hein, puisqu'il y a aussi des toitures liés à liés à l'industrie sur lequel pour l'instant, il y a pas d'obligation de désamiantage mais on sait que ça a des conséquences environnementales importantes liées notamment à l'amiante qu'on peut retrouver dans l'eau et avec avec l'érosion, donc on a vraiment nécessité d'avancer justement sur le le désamiantage et que la question du photovoltaïque en lien justement avec ses avantages plutôt intéressante puisque ça amène une une plus-Value et donc on se dit que dans le cas de ce de ce rapport, cette demande de rapport qui est plutôt intéressant qu'il serait peut être intéressant justement aussi d'avoir ce recensement parce que c'est vrai que ça soit à l'échelle à l'échelle le communal mais nos notamment à l'échelle des des syndicats d'énergie au niveau départementaux, ça serait intéressant d'avoir cette cette connaissance là pour ensuite ben permettre des dispositifs qui permettront justement de remplacer ces toitures amiantés par des des toitures photovoltaïques merci. je sais pas ce que nous dire la Ministre mais ça me paraît compliqué aujourd'hui d'enfin je ne suis pas sûr qu'on dispose des outils pour faire cet inventaire, il faudra sans doute trouver les moyens effectivement de de le faire, mais à ce stade l'imposer de cette façon-là, au travers d'un d'un rapport, ça me paraît compliqué. Donc un avis défavorable du coup pourra réfléchir et c'est plutôt pour orienter sur cette réflexion, parce que je pense qu'il faut qu'on avance sur cette question des des toitures amiantés et que le lien avec le photovoltaïque me paraît important. Donc je soumets au Sénat, l'amendement 273 avec 2 amis défavorable qui est pour.

réussite, c'est un vote et pas un débat si vous voulez bien. quels sont ceux qui sont contre. Est pas adopté. Et donc nous votons sur le onze, une nièce dans son ensemble qui est pour. Contre il est adopté, après cet article onze nièce, nous avons un amendement portant à 10 articles additionnels de monsieur Gremillet qui prend la parole. Oui merci monsieur le président, Mesdames, Nice, monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement a pour but de toute simplement d'être dans la phase concrète on veut protéger les surfaces agricoles, on sait que sur les territoires, et notamment l'agriculture consomme aussi de l'énergie et notamment de l'électricité et et l'idée de faire deux à travers le remplacement notamment de ces plaques amiantés sur les bâtiments agricoles d'une opération 3 coups : pourquoi la première, c'est effectivement régler leurs problèmes de santé qui se pose un 2ème problème qui est celui de la performance énergétique puisque l'agriculture, les agriculteurs vont devoir faire des investissements sur l'amélioration de la performance énergétique de leurs bâti et puis la 3ème, c'est effectivement de produire sur ces mêmes bâtiments une production électrique à partir de photovoltaïque. L'avis de la commission sur un portable, oui. Nous avons adopté un amendement précédemment sur sur la même thématique, donc je, je, je comprends la position du de l'auteur de l'amendement, je note cependant que le dispositif proposé et peu normatif, il est simplement précisé que l'État favorise des avantages des toits des bâtiments agricoles, l'amendement ne dit pas comment et avec quels financements, donc c'est un avis défavorable je pense que le rapport permettra de d'intégrer également ces éléments. Madame le Ministre de l'avis du gouvernement.

il n'existe pas aujourd'hui de barrières législatives ou réglementaires déjà montage des toits de bâtiments agricoles ou à l'installation de panneaux photovoltaïques et donc cette expérimentation, c'est pas très bien où elle nous mène, si ce n'est peut être pour trouver des justifications un soutien financier public.

pour des raisons qui sont liées à la santé publique et puis au développement des ENR, puisque c'est le sujet du texte, je pense que cet amendement de monsieur Grimm est tout à fait volontaire votre volontariste et que pendant le temps de la navette, pardon pour la commission du développement durable, je suivrai pas pour pour ce de cette fois-ci son avis, il me semble que nous devons être volontariste sur ces 2 sujets et que, charge à nous pendant la navette de trouver les les voies et moyens pour le rendre plus opérationnel et plus opposable cher rapporteur Mandelli. Donc nous devons nous prononcer sur cet amendement 488 qui a fait l'objet de 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Et un qui est contre. Et il est adopté. Toujours en article additionnel nous avons l'amendement 269 présentée par le président Gontard, qui prend la parole. Oui, merci, merci Monsieur le Président, c'est un amendement qui a, qui a déjà été été voté ici je crois dans la dans la loi climat et qui s'adresse à la à la commande publique, notamment sur l'achat, dispositif de production des d'énergie solaire et qui veut faire en sorte qu'on intègre l'empreinte carbone et environnemental tout au long de le du processus de fabrication de l'utilisation ainsi que la valorisation après leur leur fin de vie, ça me paraît un dispositif important en tout cas, que ça soit inscrit dans la loi qui est l'obligation de mettre ces critères-là dans les a dans les alors je sais que c'est déjà possible, évidemment que je pense que c'est encore mieux si on le dit, si on l'inscrit et si on fait en sorte que ça puisse être une une réalité, je ne reviendrai pas sur les discussions que nous avons eu tout à l'heure sur la la filière et la mise en place d'une filière photovoltaïque à l'échelle de notre pays à l'échelle européenne, et que si on veut que cette filière se mettent en place, on a besoin justement de bah de prioriser d'orienter et de prendre justement le cycle de vie entier des produits qu'on qu'on fabrique et notamment l'impact carbone l'impact environnemental et l'impact évidemment social, donc ça me paraît important je redonne l'exemple que j'avais pu donner tout à l'heure sur Photowatt qui met des panneaux mais des panneaux solaires 26000 panneaux solaires qui ne choisit pas sa filiale parce que justement elle n'a pas intégré ces critères, en tout cas suffisamment dans sa commande dans sa commande publique, donc je pense qu'il a réellement cette nécessité de pouvoir l'inscrire dans la loi, merci. monsieur le rapporteur, en faire une priorité sur un certain nombre de de sujet et donc cet amendement, il me semble satisfait par le droit en vigueur et je rappelle notamment que la loi climat et résilience à renforcer la prise en compte des critères environnementaux dans la commande publique et que ces nouvelles dispositions pour naturellement bénéficier à l'achat de panneaux photovoltaïque, de la même façon, il ne sont pas nécessaire d'aller au-delà, c'est déjà intégré, on pourrait le faire systématiquement, je pense que ce qui est vrai pour les panneaux photovoltaïques l'est aussi pour pour les véhicules, moi je préférerais effectivement que la commande publique soit orienté, si possible à 100 % cent vers des produits fabriqués en France, évidemment le le le droit actuel permet d'aller assez loin je pense que c'est voilà donc c'est un avis défavorable. Madame le Ministre. Hé bien, ce sera un avis favorable, d'abord parce que nous avons ces dernières années. Qui est de reconstruire un code des marchés publics qui soit plus plus accessible, plus accessible aux PME qui tienne mieux en compte l'empreinte environnementale et et l'empreinte sociale de notre commande publique que la commande publique, c'est un outil stratégique aussi de politique économique et que je vois difficilement comment on peut s'opposer à ça, après il faudra regarder dans le détail de la rédaction du texte pour éviter de marcher sur d'autres formes de droits, je veux redire ici à monsieur le rapporteur, vous avez complètement raison : la loi climat résilience fait un pas dans ce sens là, mais laisse 5 ans pour mettre des clauses environnementales systématique de mémoire, Là on le fait sur les panneaux photovoltaïques, on a quand même un jeu d'hypothèses qui permet d'apprécier les critères qui peuvent être appliquées, il faut que ce soit des critères les plus objective able possible pour protéger l'acheteur et effectivement c'est utile d'avoir l'appui d'experts comme l'Ademe qui aide à construire ses critères, mais je pense qu'on a un niveau de maturité qui est pas forcément acquis sur d'autres champs de la commande publique quand on veut trouver le bon critère environnemental.

c'est pas la même chose, c'est effectivement n'espérez que toutes ces ces critères loi soient pris sur l'ensemble des, des, des marchés publics, je pense que là on a c'était porte opportunité sur la question du photovoltaïque et sur une question quand même qui est important de sur cette question du photovoltaïque, même quand on parle d'acceptabilité, si à un moment donné on développe du photovoltaïque, mais effectivement qui vient intégralement Chine, je pense qu'on va avoir vraiment un problème d'acceptation sur notre sur nos territoires, donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur cette question là, là, il me semble qu'on a un levier qui est intéressant qu'il est important qu'effectivement de la musique, il faut être le retravailler le discuter, ça je suis tout à fait prêt à en discuter, mais il me semble que c'est un signal important est important sur justement cette filière photovoltaïque. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, on va soutenir cet amendement. Madame la ministre a raison, la commande publique est importante si on veut développer et structurer la filière, puis il y a une petite contradiction à droite. Je la pointe. Avec amitié, Monsieur le Président, Karoutchi tout à l'heure, on a une prise de position forte en me disant que développent les ENR ne développe les vénère, c'est le marché chinois qui va être content, Dans la commande publique. Des entreprises et des filières, les structures en France et ce que je j'ai j'ai un peu de mal ce le rapporteur à comprendre pourquoi vous refusez cet amendement. On ne peut pas avoir le discours tout à l'heure et puis quand vous propose de de soutenir pour équilibrer les choses et pour soutenir. De produire en France sur cette question là comme sur beaucoup de choses et on a un vrai débat sur la reproduire en France notamment, et le prof le plan France 2030, que vous ne soupçonniez pas cet amendement, donc je propose que, enfin, nous, nous nous sommes d'accord et nous le redisons, on pense qu'il a un gros manque sur ce texte, c'est notamment la filière industrielle, les savoir-faire donc très bon amendement et j'espère que nous serons nombreux et nombreux à le voter.

la législation existante, répondre à la demande de l'amendement ou que, effectivement, la position du du du du du gouvernement soit avéré, il n'en reste pas moins que moi, je m'interroge les les outils qui sont à disposition des des acheteurs pour intégrer les analyses un cycle de vie des produits susceptibles d'être d'être je pense que, aujourd'hui, on est très dépourvu en la matière, Madame la Ministre là a effleuré le le sujet dans son intervention, c'est c'est très pratico-pratique donc ma ma ma question, Madame la Ministre, si si, vous pouvez y répondre c'est comment allez vous développer ces informations, ces méthodes pour qu'effectivement de manière très basiques, les acheteurs puissent se référer dans leurs critères d'achat, les analyses un cycle de vie des, des, des, des produits, objets de de marchés publics. Entendu, monsieur le rapporteur souhaite s'exprimer à nouveau. Oui, j'en j'en, j'entends bien, tous les arguments qui ont été développés, je les partage à la fois parce qu'en tant qu'élu local, quelques fois, j'ai eu des remarques de la Cour des comptes parce que je ne respectaient pas le code des marchés publics pour favoriser entre guillemets avec des de vie différent et cetera et des productions locales plutôt que d'autres, dans tous les domaines, donc j'ai entendu ce que vous avez dit madame la Ministre, effectivement, il faut des marqueurs et des symboles, même si c'est déjà satisfait en grande partie, moi je propose à la Commission facilement de la commission sont d'accord, de changer mon avis de donner un avis. Favorable à une condition pour pourquoi uniquement les panneaux photovoltaïques et, pourquoi pas, toutes les autres sources ou produits destinés à produire des des énergies renouvelables, on a des fabricants en France, j'en connais en Vendée important qui un leader national sur des produits, je vais pas le citer, moi je serais très heureux que dans la commande publique, on puisse favoriser les produits fabriqués dans tels ou tels départements mais sur des critères environnementaux, évidemment non, non, mais sur l'analyse du cycle de ville mais je je partage, mais voilà, mais on peut s'en tenir au photovoltaïque, mais ayons une réflexion plus large. Oui monsieur Gremillet avait demandé la parole oui. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais remercier notre rapporteur. Parce qu'effectivement il vient prolonger le travail du Sénat, souvenons-nous, et je le dis parce que, à l'époque j'étais rapporteur sur le texte et Madame la Ministre. Madame la Ministre. Madame la Ministre je, je suis vraiment heureux d'avoir entendu votre propos tout à l'heure. J'ai encore en mémoire et pour celles et ceux qui étaient présents dans l'hémicycle à l'époque, les débats que nous avons eu pour obtenir qu'on fasse, qu'on prenne en compte le bilan carbone. moi je soutiens effectivement cet amendement, je reste cohérent, je me réjouis qu'on aille un peu plus vite que ce qu'on a été capable de faire voter à l'époque, mais quand je j'ai encore en mémoire, c'est le Sénat qui a introduit cette notion de bilan carbone et je rejoins notre rapporteur le bilan. Le bilan carbone, il ne s'arrête pas au photovoltaïque, la notion de bilan carbone, elle doit être intégré, y compris sur la c'était l'esprit du vote qui a été fait au niveau du sénat à l'époque, on ne peut pas d'un côté à avoir un discours sur le renouvelable sur l'atteinte des objectifs de neutralité carbone en 2050 et et d'être complètement incohérent par rapport au reste sur la mesure de l'impact carbone des choix que nous faisons, on est en train de légiférer, moi je me réjouis de la position de notre rapporteur parce qu'effectivement il projette dans le futur, une notion chère au Sénat qui a été très offensifs sur cette notion de bilan carbone et nous soutenons enfin je soutiens nous soutenons cet amendement. Oui, à mon tour, je voudrais insister sur l'importance du bilan carbone est en effet pas seulement dans le photovoltaïque, mais on sait que dans le photovoltaïque, il y a quelques exemples récents qui nous convainc que quand même il y avait moyen de faire quand EDF choisi des alors, c'est une de ses filiales Photowatt choisi d'acheter en Chine, vous allez pas me dire que par un peu d'astuce juridique et technologique, on aurait pas pu choisir par quel miracle, quand vous regardez les autres pays européens sur l'ensemble de leurs achats publics, ils ont massivement des achats venant de leur pays quand il y a la technologie dans leur pays, le comble étant quand même l'agriculture ou dans les cantines allemande on mange massivement allemand tandis que dans les cantines françaises la pénétration, de le des importations sont considérables, mais passons dans cette affaire il faut est la question du bilan carbone et un travail de filière, moi j'ai vu au Parlement européen, comment travaillait nous homologues des autres pays ils unissent par filière leurs chercheurs leur usine leurs entreprises productrices, parfois même les consommateurs ou les associations écologiques et il définit des priorités de Free lierre, des critères technologiques considéré comme bon et après dans l'appel d'offres et ben vous introduisez des critères de qualité des critères technologiques éventuelle adossée à la performance environnementale et carbone, donc non seulement il faut changer notre organisation des marchés publics, on est plus royaliste que le roi dans la dans la libre concurrence sans prendre en compte cette dimension vitale de notre avenir industriel et par ailleurs réellement structuré des filières avec l'ensemble des partenaires et acteurs de la filière pour qu'elles évoluent avec les critères qu'on mettra en oeuvre dans notre développement économique et nos marchés publics soient priorité soit prioriser vers la production française. Madame la Ministre. à la base pour qu'après produit soit acheté, il faut qu'ils soient de qualité et que son bilan soit positif, donc de jeu comme il y a eu des exemples qui ont été cités, je me permets de le dire, la 2ème chose c'est qu'aujourd'hui on n'a pas forcément des analyses cycle de vie complète, vous le savez, d'ailleurs c'était la question très juste, que vous avez posé monsieur le sénateur, en revanche, on commence à avoir une certaine maturité sur certains critères, je pense que sur les éoliennes terrestres les éoliennes marines et les panneaux photovoltaïques, c'est un travail qui a y compris été fait avec au niveau européen, on s'est posé la question de sur les batteries électriques aussi, on a ces éléments-là du contenu carbone et cetera de qu'est ce que peut être la bonne approche le bon critère pour justement protéger les les acheteurs parce que vous l'avez très bien dit monsieur le rapporteur, c'est pas le tout d'avoir cette approche là dans les contrats, encore faut-il ne pas se retrouver devant le juge à devoir s'expliquer d'avoir pris le mieux disant, et pas le moins dix ans et donc ça c'est un travail qui reste à mais il me semble que on a on pourra travailler dans le dans les jours qui viennent, et puis c'est aussi un travail réglementaire que on a aujourd'hui un niveau de maturité raisonnables pour faire éoliennes marines éolienne terrestre et photovoltaïques et batteries électriques, c'est pas vrai de tous les marchés de tous les dispositifs Monsieur Dantec, demande la parole aussi sources de production électrique qui sont l'éolien et le nucléaire, là il y a des filières en France mais on a un retard spécifique sur le photovoltaïque qui justifie effectivement qu'on dise on ne on a besoin maintenant d'organiser une une filière et d'amener donc le code des marchés publics jusqu'au maximum et Madame, le ministre a raison de rappeler que si ce sont des critères environnementaux, il faut être production française soit concurrentiel. Donc je mets aux voix l'amendement 269 qui fait l'objet d'un avis devenu favorable de la commission est également favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Bien. Il est donc adopté et j'imagine que d'ici sur l'aboutissement, il vaudrait mieux qu'il atterrisse dans le code de la commande publique plutôt que dans celui de l'environnement. Nous passons à la l'amendement 348 présenté par Madame de Marco. Merci monsieur le président, madame la ministre, hé bien, cet amendement est complémentaire à celui qui vient d'être voté, comme nous l'avons vu la production de panneaux photovoltaïques et, pour l'essentiel, localisée en Chine et des filières de production française et européenne qu'on commence à se construire avec le déploiement par exemple des parcs photovoltaïques le 1er parc photovoltaïque de France se situe d'ailleurs en Nouvelle Aquitaine en 2020 heure d'électricité ont été produites couvrant 9 % de la consommation annuelle d'électricité de la région en Gironde monsieur le rapporteur, la cité tout à l'heure, il y a une usine qui recycle actuellement des panneaux photovoltaïques à Saint-Loup baisse une filière d'avenir qu'il faut également encouragés à se développer sur une logique de circuits courts pour réduire au maximum l'empreinte environnementale de toute la chaîne de production, cet amendement vise donc à encourager le développement de filières de proximité pour réduire l'impact environnemental des importations et développer les circuits courts en prévoyant qu'au moment des appels d'offres, ce critère rentrent en compte pour déterminer l'attribution. la commission. Oui, c'est cet amendement pour nous, est satisfait puisque la creux intègrent déjà des critères environnementaux dans ces appels d'offres, cet amendement donc recevra un avis défavorable. L'avis du gouvernement. Favorable par logique par rapport favorable. Nous pouvons donc nous prononcer sur cet amendement 348 qui fait l'objet d'un avis défavorable. De la commission est favorable du gouvernement qui est pour.

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, cet article intègre in extenso la proposition de loi pour un développement raisonné de l'agrivoltaïsme loi dont l'objectif est de poser un cadre juridique et budgétaire cette filière en pleine expansion, nous soutenons le principe de ces dispositions, poser un cadre, même s'il est perfectible, est nécessaire et attendue par les acteurs sur le terrain, nous ne reviendrons pas sur l'ensemble des points qui ont déjà fait débat il y a à peine 2 semaines nous avons souhaité malgré tout déposé quelques amendements et c'est pour ça que je prends la parole qui pour nous sont nécessaires afin de border au mieux le dispositif global pour la préservation du foncier agricole car c'est un point central et a apporté une définition réellement protectrice pour les agriculteurs pour leurs revenus et leur production agricole malgré les débats antérieurs qui ont déjà eu lieu plusieurs points posent encore question notamment sur le risque de spéculation foncière et les problèmes de transmission qui peuvent en découler, dans un contexte de doublement des prix des Terres agricoles en 20 ans dans un contexte où le renouvellement des générations agricole s'impose comme un défi majeur, il faut également éviter à tout prix duty d'utiliser la production agricole comme un alibi au profit d'une production énergétique plus rentable, un colloque a été organisé sur ce sujet il y a 2 semaines, également, il a réuni de nombreux acteurs du monde agricole et de l'énergie, l'idée d'une convention tripartite entre le propriétaire, l'exploitant et l'énergéticien a été posée. Si la disposition n'est pas encore mûr, il est clair qu'associer l'ensemble des parties prenantes pour élaborer ensemble la pertinence du projet nous paraît non seulement nécessaire et utile, mais elle semble indispensable pour avoir une réelle acceptabilité par l'ensemble du monde agricole, merci. monsieur le président, vice-mes chers collègues, comme je suis un peu teigne, je reviens sur mon intervention d'hier matin en discussion générale comme vous le savez l'intégration au projet de loi par voie d'amendement de la proposition de loi relative au développement raisonné de l'agrivoltaïsme, récemment votée au Sénat et cohérente au regard des enjeux que présente l'installation d'équipements de production d'énergie solaire en zone agricole, ces installations sont donc amenés à se multiplier dans les prochaines années sur notre territoire, il convient donc d'être très vigilants quant à la préservation du foncier agricole et des risques de spéculation moins Tarzan concerne essentiellement donc l'amendement déposé par notre collègue Nathalie Delattre qui à permettre aux exploitations agricoles à vocation pédagogique, d'ailleurs j'ai entendu des des remarques de soutien hier matin qui sont gérés par des établissements publics ou privés sous contrat de formation agricole de bénéficier du régime de soutien spécifique à l'agrivoltaïsme, les fermes pédagogiques exercent des missions essentielles de formation aux réalités de l'exercice du métier d'agriculteur et aussi de ses évolutions et la mise en place d'installation agrivoltaïsme sur leur exploitation agricole future, elle peut pleinement participer à ces missions cette intégration nécessaire puisque telle que rédigée l'article 11 des siestes exige la présence d'un agriculteur actif et c'est le cas cependant, cet amendement de notre collègue a été déclarée irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, pourtant, il ne pouvait pas créer plus de charges publiques que l'intégration de la promotion de l'eau elle-même qui a pu outrepasser le filtre de la recevabilité financière, alors j'espère, Madame la Ministre, que vous soutiendrez l'intégration des fermes pédagogiques au sein du dispositif spécifique prévue par l'article 11 des sièges de ce projet de loi. Merci, monsieur le rapporteur, vous souhaitez également. Parlé en introduction de l'article, merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues peut être dire et redire ce que j'ai pu évoquer en commission et dans la discussion générale que dans l'esprit, nous avons amené l'agrivoltaïsme parce que c'est une, c'est une façon de faire de d'énergies renouvelables et comme ça venait de passer au Sénat il y a quelques jours, il ne semblait bon de l'intégrer dans la loi, ceci étant de pas refaire le débat j'aperçois pas Franck Monod Monod villes qui était rapporteur puisqu'on retrouve les mêmes amendements de quelque chose qu'on vient de voter, il y a quelques jours, donc c'est une question de cohérence, c'est pour ça que ça nous amène à mettre des avis défavorable aux amendements puisque l'esprit de l'agrivoltaïsme dans la loi, développement des énergies renouvelables, c'est bien d'inscrire l'agrivoltaïsme dans cette loi là et mais pas refaire le débat que nous avons eu, il y a quelques jours et et vous rappelez, et c'est heureux, puisque c'est sorti du Sénat, que ça a été voté à une très large majorité, puisque c'était 251 pour et 3 contre voilà en souci de cohérence pas refaire le débat et de pas reposé les mêmes questions qui ont été votées il y a quelques jours, voilà, je voulais faire ce petit propos là avant de démarrer. Utiles conseils donc nous commençons avec l'amendement 216 présenté par Messieurs Moga, qui prend la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le texte issu de la commission prévoit d'insérer au sein des grandes priorités de la politique énergétique française, l'objectif d'encourager la production d'électricité issue d'installations voltaïque or. Dans l'article du code de l'énergie qui définissait priorité il est fait aucune mention de l'éolien terrestre ni même du photovoltaïque, la vision de l'agrivoltaïsme, porté par la filière agricole, insiste : avant toute chose, sur le principe de symbiose entre l'activité agricole et la présence des installations voltaïque inscrire une telle objectif de production d'électricité issue de l'agrivoltaïsme, alors même que le photovoltaïque classique n'y figure pas pose un problème de hiérarchie des priorités, cet argument est d'autant plus valable que le texte voté en commission, prévoit des mesures d'équipement obligatoire de l'équivalent de 7 à 11 gigawatts de parking ombrière photovoltaïque et en définitive, c'est Thomas demande que je vous présente présente et qui est soutenu par mon collègue Longeau avec qui nous avons fait une PPR sur l'agrivoltaïsme proposent donc d'inscrire comme objectif de la politique énergétique française d'encourager la production d'électricité issue en priorité d'installations photovoltaïques implantés sur des surfaces artificialisées au sens du cours de de l'urbanisme, c'est-à-dire les parkings et hangars les toitures, les bords de routes, de voies ferrées etc, cette position est fortement par âgé partagé pardon avec le monde agricole. En discussion commune, nous devons aussi examiner le 487 présenté par Monsieur Gremillet, qui a la parole. Oui merci monsieur le président, un ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, j'ai bien entendu votre propos sur la rapporteur. La proposition que je fais à travers cet amendement et la prolongation du débat que nous avons eu sur le texte agrivoltaïsme je parle sous le contrôle de celles et ceux qui étaient présents du débat que nous venons d'avoir, à l'instant et effectivement je de dire que la profession agricole et est très attentive à cette production d'énergie renouvelable et notamment à partir du du photovoltaïque et que, en droite ligne de ce qui a été voté tout à l'heure de remplacer lorsque nous avons des toits amiantés c'est toits amiantés par des panneaux photovoltaïques, donc c'est le prolongement de l'amendement qui a été voté tout à l'heure au niveau de cette séance.

Oui, merci Monsieur le Président, je vais faire un un propos liminaire, qu'il explicitera ma position sur les amendements à venir, je veux d'abord saluer le travail qui a été fait pour aboutir à une proposition de loi au Sénat sur l'agrivoltaïsme, qui permet, je crois, de manière très consensuelle de reprendre ses textes dans le projet de loi, énergies renouvelables, vous savez que le président de la République et le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et ce n'est pas neutre dans la discussion que nous avons était favorable à à c'est que un chapitre figure dans la loi, ça c'est le 1er élément le 2ème élément, c'est qu'on a évidemment bien en tête cet équilibre qu'il faut savoir trouver entre souveraineté alimentaire et et souveraineté énergétique, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette position, c'est-à-dire que la souveraineté alimentaire, elle doit être à tout prix préserver, et on voit la fragilité aujourd'hui de cet enjeu avec la la guerre en Ukraine et la pression sur les engrais et sur les exportations. On ira aussi à l'Assemblée nationale sur neige ou sur une régulation du photovoltaïque sur les sols agricoles il s'agit pas d'en mettre partout, il s'agit bien d'avoir une vision avec des installations démontables, des installations qui permettent les cultures des installations qui sont conciliables avec la politique agricole commune et il ne s'agit pas de transformer nos agriculteurs en énergéticien je pense que ces ces points sont sont acquis dans le droit fil des débats que vous aviez déjà eu, je vais pas refaire ces débats là mon collègue Marc Fesneau étaient présents au banc, donc j'aurai beaucoup d'amendements beaucoup de d'opposition demande de retrait satisfait au retrait ou défavorables peut-être quelques avis de sagesse lorsqu'il s'agit de de rédaction, voilà ce que je voulais préciser donc au cas d'espèce, c'est un avis défavorable. Sur les deux alors nous avons le président Longeau, qui demande la parole sur un de ces 2 à ces deux amendements. la PPL qui a été voté, comme l'a dit le rapporteur il y a 15 jours, et je pense que c'est important et on va peut-être pas refaire le débat c'est c'est c'est important qu'elle a été intégrée et je remercie la commission d'affaires économiques le le rapporteur de de l'avoir fait, je crois qu'il y a eu un un bon débat il y a déjà eu un débat quand on a présenté avec Jean-Pierre Moga la la la, PPR et la APP, elle a fait la suite de de de pour ne pas trop retarder le le le débat, je crois qu'il y a des et les les éléments ont été dit au moment de la de la PPL merci. Donc nous allons nous prononcer sur ces deux amendements qui font l'objet de 2 à, de 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement, d'abord le 216 de messieurs Moga, qui est pour.

de rendre, et notamment ces plaques au niveau des bâtiments d'élevage et et Madame la Ministre soyez attentive à ce qui se passe au niveau communautaire. Je ne suis pas dans tous les secrets, mais il n'empêche qu'il y a une petite onde qui est en train de circuler sur la mise en conformité et l'obligation pour tous les bâtiments d'élevage, il y a des animaux présents d'une politique de désherbant tirage donc c'était peut-être quelque part d'être un peu avant-gardiste sur le sujet, je suis heureux et je voudrais remercier ensemble de mes collègues sur le vote que nous avons fait tout à l'heure parce que ça permettra effectivement de remplir 3 missions donc compte tenu que le cet amendement a été voté tout à l'heure, j'en suis très satisfait et j'aurais souhaité qu'il soit confortée à cet instant, ça n'apporte rien de plus, je vais le retirer mais j'aurais préféré que notre rapporteur s'adapte au vote qui était intervenu heure dans l'hémicycle il est retiré, compte tenu du vote précédent.

Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur effectivement. Ce ce. Sujet a déjà été traité il y a une quinzaine de jours mais je vous rappelle qu'il

et sénateurs socialistes maintiennent la position qui avait été la leur lors de les débats sur la PPL nous souhaitons donc encadrer davantage le texte actuel pour éviter toute dérive, comme l'a évoqué, Madame la Ministre, vers un modèle énergie culture pour cet amendement, nous proposons de renforcer l'ambition du texte en prévoyant qu'il faudra remplir au moins 2 des services qui sont cités dans le texte donc dans cette optique, remplir donc de service ne nous sommes pas insurmontable, voilà quelle est notre proposition. Dans l'ordre qui est prévu, c'est ensuite l'amendement 231 de monsieur Cabanel, qui a la parole. recommandations par rapport au débat que nous avons déjà eu mais rien ne m'empêche quand même de dire que je suis quand même assez craintif, par rapport à la définition qui avait été voté ici au Sénat, qui à mon sens ne nous protégera pas suffisamment des projets dits alibi, ça a été évoqué et Madame la Ministre, vous le savez, à terme, donc de rapport de gay pour éventuellement l'agriculteur il y a pas photo entre la production d'énergie et la production agricole et c'est là que, il va falloir quand même savoir où on va mettre le curseur parce que j'ai peur qu'il y ait des dérives et comme vous l'avez souligné il faut il faut effectivement abordé ce sujet dans sa transversalité hein tant que souveraineté énergétique mais aussi souveraineté alimentaire.

et, et, donc, dans le prolongement de ce qui vient d'être évoqué, il s'agit pour nous de veiller à ce que l'activité cette activité ne devienne pas le prétexte activité l'agrivoltaïsme ne devienne pas le prétexte à une production d'énergie, même si cette dernière est est renouvelable à vertueuse est, qui s'inscrit dans les objectifs nationaux et européens de développement des ENR c'est pourquoi dans dans le cadre du futur décret donc qui mettra en oeuvre cette loi, la production agricole et les revenus qui a son tissu doivent rester prépondérant, une fois de plus là lors des débats sur l'APP à l'agrivoltaïsme le la réponse qui nous a été apportée n'était pas clair donc je peux toujours espérer qu'elle soit clarifiée aujourd'hui le rapporteur, vous avez indiqué que notre abonnement était redondant avec les définitions déjà retenue, tout en précisant également qu'il reviendrait à exclure de la définition des agriculteurs pouvant rencontrer des difficultés ponctuelles de production ou de revenus, ce qui, malheureusement, est le cas aujourd'hui de bon nombre d'entre eux, donc il faudrait savoir soit notre amendement est satisfait, soit il modifie la portée du texte, en tout état de cause, nous maintenons notre position, à savoir l'activité agricole et les revenus qui en sont tirées doivent rester le moteur d'une exploitation agricole. De l'université. Donc maintenant il me faut, il nous faut l'avis du rapporteur sur les deux amendements 507 et 509. Merci, merci Monsieur le Président merci à mes collègues pour leur compréhension, j'aurai toujours la même position, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable.

tout va se passer à ce niveau là, même si notre notre assemblée abordé le sujet avec les 4 critères et et et des critères aussi complémentaires,

comment envisagez-vous cette phase-là, parce qu'encore une fois, elle nous intéresse tous et et et et elle va, elle donnera in fine et la la la la définition et les possibilités en la matière, je vous remercie. Donc nous allons nous prononcer sur pardon Monsieur Melville. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je suis un peu surpris par les les inquiétudes que suscite ce développement de l'agrivoltaïsme surtout, on avait commencé à travailler sur la la PPA avant la crise ukrainienne, mais il y a eu, il y a eu en plus es bon évidemment dans des besoins énergétiques évident aujourd'hui, donc ça ne peut qu'améliorer notre mix il y a eu aussi beaucoup d'expérimentations sur le terrain qui ont montré dans les zones, notamment les plus touchés par le changement climatique, je pense au au Sud-Ouest au Sud-Est, les bénéfices de l'installation de de faux panneaux photovoltaïques inclinables sur le rendement des cultures sur sur les les Terres d'élevage avec de l'herbe qui repousse beaucoup mieux une limitation de de l'évaporation,

tous les voyants semblent dans le Vert, toutes les planètes semblent alignés et surtout un revenu complémentaire pour les agriculteurs, non, moi je vois pas de risque de de dérive de production énergétique alors que le critère principal, c'est le maintien de l'activité agricole et on va voir en plus une amélioration de ses rendements agricoles, or le maintien de l'activité agricole est facilement vérifiable, donc je crois qu'il ne faut pas trop se faire de soucis, on le le le le territoire français ne sera pas inondé de de panneaux photovoltaïques, puisqu'il y a quand même des des investissements, il y a tous les avis tous tous les les garde-fous qu'on a mis en place, donc j'ai du mal à comprendre toutes ces inquiétudes. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 507 de monsieur renonce Rungis qui a fait l'objet de 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Il n'est pas adopté. Et nous nous prononçons sur le 505 même vote. On raconte

Même vote, donc il est repoussé également. Nous avons maintenant l'amendement 505 de monsieur au donc sarrasin qui a la parole.

laissé au moins législateurs que nous sommes la possibilité de préciser le le le au maximum le cas général, de la loi de parce qu'aujourd'hui, de le le le décret ne nous permet pas d'y voir très clair, donc j'espère, Madame la Ministre, que dans votre avis vous répondrez à la fois donc aux aux propos de de mon collègue Montaugé et à sept avant.

Madame la Ministre, sur l'amendement 505. également avis défavorable à votre demande de retrait sinon avis défavorable et, pour répondre très rapidement, hein, comme je l'ai dit à l'Assemblée Nationale nous ferons des propositions en matière d'encadrement du photovoltaïque posé au sol il te le décret parce que c'est du réglementaire, ça, il y a pas photo, il sera pris en interministériel et avec les consultations usuel et notamment celle, s'agissant de ma filière du Conseil supérieur de l'énergie et évidemment du côté de l'agriculture, en prenant en compte les avis des des des représentants des parties prenantes, et donc je pense qu'on arrivera texte équilibré et je le redis, enfin il y a pas d'ambiguïté sur la position du gouvernement sur ce que nous souhaitons faire, je pense que nous avons une politique en matière agricole, qui est tout à fait ambitieuse et engagé. Est-ce que vous mettez l'amendement donc je mets aux voix l'amendement 505 avec un double avis défavorable qui est pour.

pas adopté l'amendement 506 du même auteur, vous avez la parole. Donc je je parle en même temps des 5 sens du 500 du 508 et ce sera ma contribution à la l'allégement du débat sur ce sujet puisque ils sont assez techniques et donc je retire ses deux amendements.

Saint-34 mais je voudrais, Madame la Ministre, vous dire que le 232 correspond et il reprend une recommandation donc de la mission d'information flash qu'il y avait eu lieu à l'Assemblée nationale portant sur l'agrivoltaïsme, donc j'espère que, lors du débat à l'Assemblée nationale, vous tiendrez compte de cette mission d'information flash pour effectivement tenir compte donc d'un partage équitable de la valeur avec la les agriculteurs.

Merci monsieur le président, madame le Ministre, celui-ci n'est n'est pas retiré, je voudrais juste revenir sur sur un point, ça concerne vraiment l'acceptabilité de l'agrivoltaïsme, ce qui fait peur aujourd'hui au monde agricole, mais aussi aux défenseurs du paysage, c'est d'avoir des nappes de plusieurs dizaines d'hectares de panneaux photovoltaïques, même s'ils sont de faible densité pour l'agrivoltaïsme, cet amendement vise à limiter ça sera sans doute définie dans le décret, mais c'est pour soit soit bien n'inscrit quelque part limitée à 1 mégawatts la puissance par exploitation, ce qui permet d'avoir une répartition assez harmonieuse sur le territoire hein mégawatts de puissance par exploitation agricole oh comme ça ça va éviter des grandes nappes et ça permet quand même d'avoir une production subséquent. J'ai rapporteur. Même avis monsieur le président, demande de retrait ou avis défavorable. Le ministre, même chose. Je mets aux voix l'amendement 323 avec double avis défavorable qui est pour.

principal doit notamment et non peut s'apprécier au regard du volume de production du niveau de revenu et de l'emprise au sol, cet amendement, donc il avait été rejetée lors de l'examen de la PPL au motif que la rédaction que nous proposions à l'époque, réduisez la précision de à, seuls 3 critères alors que d'autres pouvaient être utile, c'est pourquoi nous propose une nouvelle rédaction en en précisant notamment qui permet de s'assurer du respect de ces 3 critères sans fermer la porte à d'autres critères par cet amendement des sénateurs donc souhaite lutter contre les effets d'aubaine et mettre en place les garde-fous pour éviter que l'activité agricole ne devienne une excuse à une production d'énergie qui est une dérive qui a quand même été évoqué à plusieurs reprises par nombre de nos collègues sénateurs, donc ça veut bien dire que ce n'est pas si anodin que ça. Pas d'intervention, donc je mets aux voix l'amendement 510 faisant l'objet d'un double avis défavorable qui est pour. Et

parle plutôt de l'après, puisque il vise à mettre l'accent sur la nécessité de mettre en place un suivi et un contrôle réel des installations sujet qu'on a assez peu évoquée jusque-là afin de s'assurer du bon respect de la loi et de l'esprit qui était notamment celui du précédent autre amendement d'une manière générale, nous sommes toujours inquiets de l'adéquation entre les moyens financiers et humains mis à disposition par les services de l'État dans le cas de la mise en oeuvre une politique publique et la réalisation de l'ensemble des missions de contrôle qui sont liés c'est pourquoi toujours dans le même souci de préservation de l'activité agricole, nous souhaiterions que tout soit mis en oeuvre pour éviter qu'une installation agree voltaïque une fois autorisé ne fassent plus jamais l'objet d'un contrôle, ce qui ouvrirait la voie à des dérives certaines l'article 40 limitant fortement notre Champ d'action, nous demandons que le futur décret puisse, outre le fait de prévoir les modalités de suivi et de contrôle, évaluer les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. Donc, nous nous prononçons sur le 511 nous recomptant qui est pour.

Je vais vous demander de vous lever, qui est pour d'abord.

Eh bien il est adopté. Hé oui, avec une voix de de différence. Nous passons au 514. Monsieur le Président, Madame la Ministre, puisque nous sommes sur la bonne voie, je continue. Non, non. Donc nous abordons ici un amendement très important pour notre groupe, puisqu'il vise à prévoir une information systématique et obligatoire des maires des communes concernées par l'implantation d'une installation agree voltaïque peine à renforcer l'acceptabilité et surtout de ne pas laisser les maires devant le fait accompli concernant les projets qui pourraient avoir des nuisances pour les riverains, nous proposons donc que cette information soit assortie de la possibilité pour le maire d'émettre des observations et de sel pour le porteur de projet, il y apporter des réponses et à l'aune des débats qui nous occupe, qui nous ont occupés depuis nombre de nombreuses heures, il nous semble pas opportun de donner un pouvoir décisionnaire Omer pouvoir qui pourrait les mettent dans des situations très difficiles vis-à-vis de leurs administrés, nous estimons qu'un cadre clair soit posée pour les que les élus locaux soient également informés et donc partie prenante des décisions parfois structurantes qui sont prises sur leur territoire. L'avis de la commission. les documents procédures et délais visés pourront être spécifié cette occasion enfin dans le cadre de ce projet de loi, l'article III vu précédemment applique pour tous les projets d'énergies renouvelables et, dans le cadre des schémas de cohérence Lescott l'accord des communes et de leurs groupements, c'est donc un avis de retrait ou de un avis défavorable, Ah, du gouvernement, il satisfait donc demande de retrait. Retrait il est retiré, merci, nous passons au 218 présentée par Messieurs Moga, qui a la parole. Merci monsieur le président, je le retire. Merci, ensuite nous avons quatre amendements en discussion commune nous commençons par le 341. Qui le défend, la présidente, monsieur le rapporteur, il s'agit d'un amendement déposé par notre collègue du plomb et plusieurs autres collègues, cet amendement vise à prévoir des garanties plus précise quant à la réversibilité, aux conditions de démantèlement des installations à agricoles voltaïque, pardon, condition essentielle à l'absence d'artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols. L'amendement en discussion commune identique 389 et présentée par. Madame, il vient d'être défendu président. Et Monsieur Gremillet par le pour le 400 93. Oui, monsieur le président je vais aller très vite, puisque je vais le retirer, puisqu'hier dans les débats, il a été satisfait à la fois par le rapporteur par Madame le Ministre, donc il a il a plus d'objet merci.

merci Monsieur le Président, dans le ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à rendre automatique la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état d'un site pour les projets dans la limite de puissance installée est supérieur 1 mégawatt la rédaction actuelle qui ouvrent seulement une possibilité semble en effet peu contraignantes, à nos yeux, les sénateurs socialistes réaffirment que la remise en état d'un site agricole doit être un élément constitutif du projet gris voltaïque, il s'agit de préserver le foncier, quelle que soit la taille ou la puissance des installations qui émergeront sur les territoires, à l'heure des débats sur la préservation de notre souveraineté agricole chaque mètre carré de terre agricole doit faire l'objet d'une attention toute particulière.

Il fait l'objet d'un double avis défavorable et je le mets aux voix qui est pour. Contre. Il est pas adopté. Nous avons ensuite à nouveau 4 amendements en discussion commune le premier le 233 présenté par monsieur Cabanel. Il est retiré. Thierry nous avons ensuite hein 491 présenté par Gremillet. Compte tenu de ce qu'a dit le prix notre rapporteur monsieur le président, je le retire aussi. Tiré Monsieur Salmon. Merci monsieur le président, le ministre, je reviens sur cet amendement là parce que ça concerne l'avis conforme de la Cdpenaf concernant les projets d'agrivoltaïsme et de mémoire, il me semble que lors de la loi que nous avons examiné il y a 2 semaines, c'était passé à une ou 2 voix près, donc c'est pour ça que je me permets d'y revenir, donc j'estime que cet avis conforme est une vraie demande de plusieurs syndicats agricoles et je crois que c'est très partagée sur ces bancs, c'est aussi une demande de l'Ademe, donc voilà cet avis conforme, pourrait être très bien perçus, merci.

et donc pour rester dans la droite ligne de ce qu'a dit notre rapporteur, je retire cet amendement puisqu'il a été partiellement satisfait hier. Alors maintenant Monsieur là, le rapporteur, il nous faut l'avis sur le 321 qui reste.

je veux rappeler. Avec force, je veux rappeler à à mes à mes collègues que nous n'avions pas voter la Cdpenaf parce que ça retire le pouvoir au maire, je le répète, je le redis voilà. Quels sont ceux qui sont pour. pour. Il n'est pas adopté. Ensuite trois amendements en discussion commune le 1er émanent de notre collègue Demilly il est défendu par Me zapper à nouveau. Merci président, cet amendement vise à sécuriser les installations photovoltaïques sur les serres en gare et ombrière à usage agricole en faisant primer le projet agricole sur le projet énergétique, il s'agit de s'assurer que des bâtiments inutiles voire nuisibles à l'activité agricole ne seront pas construits uniquement pour supporter des panneaux photovoltaïques, et donc d'éviter les nombreux projets alibi notamment sous serre.

La la ministre. Alors c'est favorable sur le 388 parce qu'en fait c'est une précision utile et ses défavorable sur les autres. Je vais mettre aux voix, donc l'amendement 388 qui a un ne un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Donc, celui-là est adopté. Sur les amendements 495 et 343 ils sont maintenus.

Merci monsieur le président, c'est toujours la même : ouais, je vais le retirer pour gagner du temps, puisqu'on est à une position où effectivement on ne refait pas le débat, même si effectivement parfois il y aurait quelques précisions apportées mais je les retire les deux.

Gremillet du plaisir de défendre son amendement, je voudrais juste dire que cet amendement monsieur du plomb, complète un autre amendement prévoyant les conditions de réversibilité de démantèlement des projets qui visent à sécuriser la procédure pour effectuer les travaux de remise en état des sols. Avis de la commission. Donc 342 494. Demande de retrait ou avis défavorable. Même avis.

merci monsieur. Président Madame la Ministre, chers collègues, donc cet amendement c'est un amendement d'appel qui vise à demander la remise d'un rapport au gouvernement sur 2 problématiques importantes qui peuvent être traitées au détour cette PPL, la première c'est la nécessité d'anticiper au mieux les situations dans lesquelles un projet impliquerait plusieurs acteurs, à savoir un exploitant agricole, un propriétaire du foncier agricole, un porteur de projet d'énergie solaire tout au long des débats que nous avons vu le 20 octobre comme ceux qui nous ont occupé aujourd'hui nous avons avant tout à aborder la nécessité de préserver les agriculteurs et de ne pas détourner les Terres agricoles de leur vocation première, en conséquence, aucun projet ne doit pouvoir être menée sans concertation et accord avec toutes les parties prenantes de plus, il faut nécessairement que la répartition de la valeur ajoutée induite par la mise en place d'une installation photovoltaïque se répercute à hauteur des efforts consentis par toutes les parties prenantes, et plus particulièrement l'exploitant agricole qui sera confronté au quotidien actuellement les chartes de bonnes pratiques existent pour réguler les relations entre et encourager la complémentarité entre agriculteurs et production photovoltaïque, il faut en tirer un bilan et en fonction de celui-ci, voir si elles peuvent généraliser la seconde problématique,

déjà rappelé tout à l'heure, par ailleurs, le sujet qui nous occupe aujourd'hui nous renvoie nécessairement à des questions financières et à celle de la répartition de la fraction de la composante de l'hiver, c'est un sujet central qui captera sans aucun doute l'tension sur le terrain et il faudra nécessairement veiller à une juste répartition de celle-ci. Merci monsieur le président, j'ai juste pour vous dire que le le Sénat et par principe défavorable aux demandes de rapport et qu'il nous semble que par ailleurs le la garantie de revenus est prise en compte directement dans la définition de l'agrivoltaïsme du coup, voilà, c'était une demande de retrait ou un avis défavorable. Même avis. Bien donc je mets aux voix le 513 avec un double avis défavorable qui est

merci monsieur. Président, madame, c'est, effectivement, n'est pas normalement, mon collègue Sébastien Pla, qui vise à prévoir la la la remise chaque année d'un rapport relatif à l'impact de l'agrivoltaïsme sur le sur l'agriculture par le réseau des chambres d'agriculteurs nous estimons que l'impact des projets énergétiques sur le fonctionnement des espaces et des exploitations doit être analysée et traitée afin d'éviter une atteinte significative à la viabilité des systèmes d'exploitation, la collectivité ne dispose pas de tous les leviers sur les mutations foncière mais peut en activer certaines, notamment avec le concours de l'opérateur, tels que les affaires et bien sûr les chambres d'agriculture, la réalisation d'observatoire du foncier agricole, dont se sont dotés, certains territoires permet aussi de visualiser directement l'impact des projets urbains sur les exploitations agricoles, et en particulier donc des projets agrivoltaïsme en raison en raison des risques de captation des potentiels de Terres arables le suivi voir le réseau consulaire agricole serait une garantie pour la préservation des Terres Anja agronomique et bien sûr pour le reste allant générationnel des agriculteurs. Avis de la commission. Même chose que précédemment sur la position du Sénat par rapport au rapport, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Même même identique du gouvernement, donc le 515 avec double avis défavorable qui est pour. pour. Il n'est pas adopté, donc nous pouvons voter sur l'article onze des sièges dans son ensemble qui est pour.

Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, depuis la libération du marché de l'énergie en 2007 plusieurs fournisseurs d'énergie, dit à l'alternatif en contribué à développer l'offre d'énergie verte, ils ont aussi participé avec leurs clients au développement d'énergies renouvelables sur le territoire en offrant comme garantie de ne pas recourir à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement n'a protégé que les clients des fournisseurs historiques la crise énergétique que nous traversons, a frappé de plein fouet ces nouveaux acteurs de la transition, qui se sont trouvés face à face à un dilemme : soit préservé leur engagements commerciaux de ne pas recourir aux tarifs réglementés soit rompre les engagements commerciaux et recourir à l'énergie nucléaire. On estime aujourd'hui que 100000 clients par mois rejoignent EDF pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire ses clients de fournisseurs alternatifs semble avoir oublié avoir été oubliés par le gouvernement au moment de la gestion de la crise, ils sont pourtant les précurseurs de la transition énergétique que nous appelons aujourd'hui ne nous veut. à long terme ce précédent pourrait avoir un impact négatif sur le déploiement d'une offre d'énergie verte si rien n'est fait pour rétablir la confiance des consommateurs dans ses offres alternatives à l'énergie nucléaire. Nous avons proposé la création d'un fonds d'indemnisation pour les clients de fournisseurs qui ont vu leur facture sensiblement augmenté durant la crise notre amendement a été déclarée irrecevable, cet amendement-là vise, lui, a précisé le code de la consommation à la lumière de notre expérience, cette crise énergétique afin de renforcer l'information aux consommateurs. qu'est l'avis de la commission sur cet amendement 365 monsieur Armand. Merci monsieur le président, la mention de la proportion des énergies renouvelables dans les contrats de fourniture n'est pas souhaitable tout d'abord, il existe déjà des obligations d'information et des garanties d'origine, de plus, la neutralité technologique n'est pas respectée puisque seule la production solaire ou éolienne d'une part, ou celle de biogaz, d'autre part serait prévu, c'est donc une demande de retrait soit un avis défavorable, c'est un avis favorable bien. Je vais mettre aux voix cet amendement 365 avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement, quels sont ceux qui sont pour. Ah pardon, monsieur Guy demandé la parole pour s'exprimer. Excusez-moi, monsieur le président, je le la même et je vous, je vous remercie, non nous on soutiendra pas cet amendement. Je le dis tranquillement mais bah oui, enfin bon quand même sur la reine, parce qu'au bout du bourg, il y a une chose qu'on ne on ne parle pas là tous les acteurs alternatifs, je suis en train d'éplucher la liste là depuis des longues semaines. Quasiment tous, ils disent énergie verte. Production hydraulique, production à éoliennes et après il y a la question des certificats d'origine. D'ailleurs, là aussi, on en parle pas grand sujet. Il faudrait mettre sur la table parce que peu de consommatrices et de consommateurs savent que d'abord tous les acteurs alternatifs qui se dise vers son biberonné à la reine, alors là, avec la crise, même ceux qui avaient juré au grand coeur qui le ferait pas comme un air ils y vont. et puis après il y a tous les abus qui sont en train de se faire assez nombreux et puis il y a une dernière chose. C'est que vous pouvez avoir, dire que vous êtes Vert mais en réalité, ne faire que de la reine et que du nucléaire et après vous allez sur un autre marché acheter des certificats d'origine, il y aurait un petit débat à faire là sur les ENR, moi je suis d'accord production mais en même temps on vend le certificat d'origine faut abolir ce double marché ou on fait Croire au client qu'ils ont de l'énergie renouvelable, alors que, de toute façon tout le tout est dans le même tuyau et tout est servi par les électrons et de l'autre côté, acheter les certificats d'origine, donc je vous le dis, puisque c'est encore quelque chose pour favoriser la reine pour nous c'est vous connaissez notre position. Mais sur les certificats d'origine, on va y revenir parce que vous voulez pas en débattre, mais dans l'article 17 sur les PPA, il y aura beaucoup de choses à dire sur cette question là. Après cette explication de vote je mets aux voix donc l'amendement 365 présenté par Madame de Marco, avec un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Donc il y avait pas j'ai noté. Nous arrivons à l'article 12 sur lequel Monsieur Houlgate est inscrit. Merci monsieur le président, donc nous arrivons donc sur sur l'éolien Offshore et je vous invite mes chers collègues, à analyser cet article 12 avec une plus grande avec la plus grande prudence, je comprends que que le Sénat, chambre des territoires porte la voix des élus locaux et les élus littoraux qui se sont vu imposer des parcs éoliens, des erreurs ont sans doute été commises et et je crois que on doit l'avouer : si on avait eu à l'époque un peu de recul, nous n'aurions jamais implanté de Park aussi près des côtes, comme c'est le cas à Saint-Brieuc ah ça se

dit que les projets en mer et le raccordement font désormais l'objet d'une procédure de participation du public qui est organisée avant la désignation du développeur éolien, notamment en vue de définir la localisation, de même nous constatons aussi que que c'est ce dialogue constructif permet de trouver des consensus, donc ne rigidifie ont pas le texte de loi en nous projetant dans l'avenir, avec, peut-être, je dirais des des réminiscences du passé, même si celles-ci sont justifiées, faisons donc confiance à l'Intelligence collective car elle a fait ses preuves et et nous avons-nous trouver notamment en Manche, une zone de moindres contraintes qui satisfait tout le monde et qui se situe à 33 kilomètres des côtes, donc soyons prudents et, surtout, faisons attention à cette filière ne coupons pas les ailes à la filière éolienne marine française. Madame Breillat ça a également demandé la parole. Madame var Ayache, vous avez la parole.

Cette décision de privilégier les projets éoliens à 40 kilomètres des côtes revient à réduire considérablement les installations et pour ainsi dire à presque interdire massivement l'éolien en mer puisque tout le monde le sait : à 40 kilomètres, cela veut dire que, dans la Manche et dans la mer du Nord, il ne sera pas possible de construire des éoliennes, des éoliennes flottantes et c'est la même chose d'ailleurs en Méditerranée. Il en résulte que cette disposition consiste en fait à concentrer les éoliennes sur la façade Atlantique, notamment dans les pays de la Loire et en Bretagne, précisément, le Golfe de Gascogne, d'ailleurs, et ne parlons pas cette distance des 40 kilomètres Nous avons le devoir de veiller, c'est vrai à une juste répartition équilibrée des éoliennes marines sur notre territoire, nous savons que, précisément, dans ces territoires situés en bordure du littoral, les habitants et les élus sont inquiets et qu'il est important de le prendre en compte tant cette question tout le monde le sait préoccupe les pêcheurs Élysée et les associations de défense de la biodiversité, les dispositions résultant des votes que nous avons eues sur l'article, hein, ah et 3 redonne au maire et au conseil municipal, la possibilité d'intervenir en amont sur la validation des projets, tout comme d'ailleurs ils peuvent le faire au sein du Conseil maritime de défense dans lequel siègent les représentants des collectivités territoriales pour toutes ces raisons. Nous voterons l'amendement de suppression du gouvernement. porter trop de rigidité dans le texte par rapport à cela risque d'avoir des conséquences qui seront des conséquences totalement catastrophique et funeste pour la filière éolien Offshore je crois que c'est un élément qui est un élément partie quand même important, parce que pour une fois que nous avons une filière et qui est en train de se structurer au niveau industriel, à l'échelle nationale puisqu'on produit d'un autre pays, ces ces éoliennes pour pour la plupart par la loi impliqué un certain nombre de de d'orientation qui serait catastrophique par rapport aux perspectives de développement n'est pas une bonne chose, ensuite je crois qu'il ne faut pas souffrir de Métropolis entrisme en la matière, il faut aussi regarder les éléments par rapport à nos outre-mer et l'enjeu de développement des énergies nouvelles marines renouvelables, plus particulièrement dans nos outre-mer est un enjeu essentiel, nous avons les dernières centrales à charbon, qui sont dans nos outre-mer donc ne pas leur donner de par la loi, la capacité, la possibilité, s'ils le souhaitent, de pouvoir développer des champs éoliens, y compris plus près que 40 kilomètres des côtes serait une erreur et serait même une faute, et donc dans ce cadre-là, moi j'ai j'ai j'attire l'attention sur l'impérieuse nécessité en plus au regard de tous les éléments de concertation et qui ont été développés par les collègues et tout à l'heure de tenir compte, donc de ces cadres de spécificité, on a parlé de la Manche et de la mer du nord de la Méditerranée de la de leur situation spécifique, mais n'oublions pas nos territoires ultramarins merci. Pour essayer de faire un peu retomber la pression bon avant les votes, puisque moi je suis du Pas-de-Calais si effectivement je valide, c'est 40 kilomètres lorsque je serai invitée à poser le 1er pieux en mer d'une éolienne Offshore je suis invitée à Canterbury,

Monsieur Marchand souhaite aussi s'exprimer en préalable sur l'article. Quand le Pas-de-Calais s'exprime, il faut que le Nord prenne la relève pour dire effectivement que dans le département du Nord, on a plusieurs particularismes et d'être aussi limitrophe avec la Belgique et moi quand je vais en Belgique, et quand je vais au stand effectivement le parc éolien Offshore, vingt-trois kilomètres des côtes et visiblement, ça a l'air de ne perturber personne est quand même un élément que je voudrais amener dans le débat, alors je sais bien, comparaison n'est pas raison, mais ayons présent à l'esprit que le 19 mai dernier l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique ont ont annoncé vouloir installer pour près de 150 mégawatts d'éoliennes en mer du Nord d'ici à 2050 pour en faire la centrale électrique verte de l'Europe et se passer des hydrocarbures russes, donc je trouve qu'il serait dommageable pour des contraintes fixées de façon tout à fait arbitraire que nous passions à côté de cette belle ambition. Messieurs mais deviennent. Merci monsieur le président, dans le ministre nous dans le Sud-Ouest, ce qui nous concerne, les Anglais sont plus loin on je n'aura pas les Américains, je pense par contre gardons présent à l'esprit que ces distances de de 40 kilomètres, c'est tout simplement un enterrement du projet. Madame Saint-Pé. Oui, c'est le président, une partie de notre groupe centriste votera également pour la suppression dont votera en faveur de l'amendement du gouvernement soutiendra les différents amendements qui vont dans ce sens, considérant que, si nous n'arrivons plus à planter une éolienne en mer à moins de 40 kilomètres et que, au-delà des 40 kilomètres c'est l'éolien flottant qui aura droit de cité et que la technologie aujourd'hui n'est pas mature pour faire de l'éolien flottant, je crois qu'il nous faut prendre conscience que nous devons développer l'éolien en mer, surtout en ayant écouté, pas plus tard qu'hier soir, les informations catastrophiques d'EDF qui nous dit de voir encore repoussés l'ouverture de certaines centrales nucléaires qui sont en maintenance actuellement merci. Donc. Nous allons justement en débattre avec les 11 amendements en discussion commune nous commençons par le, 622 présentée par Madame avec. Cet amendement vise 2 choses : la première ventiler les dispositions de l'amendement initial dans les codes pertinent, tout en faisant porter le document stratégique de façade dans l'article du code de l'environnement, relatif à la planification de l'espace maritime objectif, mieux organiser la concertation, en permettant notamment pour les projets éoliens Marine un débat mutualiser sur chaque façade maritime avec les territoires et leurs habitants, le deuxième et je crois que c'est ce qui va occuper nos débats, c'est qu'il supprime la mention d'une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes en la remplaçant par la mention de l'implantation en zone économique exclusive, cette distance des 40 kilomètres des côtes et techniquement difficile à mettre en place et c'est pas moi qui le dit mais votre rapport, monsieur le rapporteur, vous écrivez que l'éolien posé ne peut être utilise que jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres, or, à l'exception de la Manche cette profondeur est atteinte à une faible distance des côtes, notamment en Méditerranée en Bretagne, en Gironde ou au large du Pays basque et il nous n'évoquons pas les territoires ultramarins qui sont les premiers à être pénalisé par cette mention, outre l'aspect technique, cela ouvrirait des sources de contentieux car les porteurs de projets devrait également prouver qu'ils ne peuvent pas le faire à plus ce seuil nous paraît donc dispo pour disproportionnée lorsque l'on sait que dans 30 % du temps, la visibilité est inférieure à 8 kilomètres pour toutes ces raisons, nous vous nous opposerons fermement à cette distance minimale de 40 kilomètres elle reviendra à inverser tout simplement l'objet de cette loi qui est, je le rappelle est d'accélérer notre production d'énergie renouvelable, je vous remercie.

sur proposition de du rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a procédé à la réécriture complète de l'article 12 du projet de loi afin d'améliorer la planification de l'éolien en mer, nous soutenons cette démarche cependant une partie de l'article propose que de nouvelles procédures de mise en concurrence et l'ancien, à compter de la publication de la loi privilégie les zones d'implantation de projets éoliens en mer situées à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes cette distance se pose des difficultés techniques, cela a été dit. Et la Commission n'en est consciente, elle peut compromettre l'éolien en mer Méditerranée, ainsi que sur une bonne partie de la façade Atlantique, certes, j'ai bien entendu, monsieur le rapporteur, ce n'est pas une interdiction d'implanter les éoliennes à moins de 40 mais quand même, cette disposition envoie un très très mauvais signal à l'industrie des énergies maritime et brouille la visibilité sur l'acceptation de leur projet, or l'aime pas paysager ne doit pas constituer le critère principal pour décider des zones d'implantation des parcs éoliens en mer alors que d'autres usages sont bien plus prioritaires tels que la pêche, le transport maritime, la défense ou la protection de la biodiversité, le prix d'un amendement vise donc à supprimer cette mesure, qui constitue un frein au développement de l'éolien en mer pour lequel la France est d'ores et déjà très très en retard. Second amendement identique Monsieur Dantec. Oui merci me monsieur le président, je crois qu'on est sur une discussion extrêmement importante et je crois aussi que, clairement, et il ne faut pas mentir aux Français, il ne faut pas mentir aux Français sur 2 points : le 1er c'est que nous ne passerons pas en termes de production électrique dans les 10, 15 prochaines années sans une production massive d'éolien Offshore, nous avons un parc nucléaire vieillissant, la dernière communication d'EDF de ces derniers jours montrent qu'on ne tiendra pas les délais, une nouvelle fois sur les rafistolages parce que là on est qu'au rafistolage, on n'est pas au grand carénage, le grand carnage dans tous les cas, va rendre une partie du parc en incapacité de production dans les sur les 10 prochaines années, donc si nous n'avons pas cette éolien Offshore, nous ne passerons pas et nous achèterons ailleurs notre électricité, ça c'est la réalité, ce sont les chiffres de RTE, ce sont les chiffres de la dame, nous le savons tous, c'est le 1er point. Le 2ème point : il ne faut pas mentir aux Français en leur faisant croire et ça a été dit avant moi par d'autres interlocuteurs par nos orateur sur le fait que nous avons des technologies matures pour expédier des parcs, très loin des côtes, ça n'est pas vrai.

ces derniers sont effectivement pas très loin des côtes est écoulé et y compris les coûts de raccordement sont un élément important du modèle économique, donc si nous voulons rester une grande nation de production d'électricité et ne pas avoir demain des électro-intensifs, soit qui achètent leur électricité ailleurs parce qu'elle sera moins cher, notamment avec l'éolien Offshore anglais, écossais, danois et de la mer du Nord en général soit avec du photovoltaïque, qui viendra du sud où là, on a du photovoltaïque, qui sort à 30 euros aujourd'hui trente euros je vous rappelle que le RPR est à cent vingt euros si on ne fait pas ça, et je voudrais juste dire que le 1er qui a mis les 50 gigawatts de de puissance sur la table, ça a été, Daniel Gremillet dans le débat de la loi climat, donc je pense qu'on a un consensus possible sur le fait qu'il nous faut, c'est 50 gigawatts pour l'avenir de la France. Merci beaucoup monsieur le président, je crois que beaucoup de choses viennent d'être exprimées et qu'effectivement, c'est une discussion qui est très importante, très importante par ce ce dont on parle, les 10 gigawatts espérer dans les 10 années qui viennent, c'est l'équivalent des 6 EPR que nous voulons lancer c'est pas rien si je perds. C'est pas rien, et effectivement, il faut reconnaître qu'un certain nombre de projets ont probablement pas. Atteint les objectifs souhaités ou que la transparence sur la visibilité sur les modalités de de construction n'a pas été suffisante comme beaucoup l'ont dit sur ces bancs déjà. On a commencé à tirer les leçons de ce là on a même tiré les leçons de cela et aujourd'hui les projets qui sont proposés sont proposées et organisé de manière beaucoup en associant beaucoup mieux les différentes parties prenantes et en faisant attention à l'impact, l'impact paysager, l'impact également je dirais en terme de conflits d'usage de ces projets et donc cette maturité, nous allons pouvoir en bénéficier dans les dans les années qui viennent. Mettre un coup d'arrêt à notre filière c'est aussi poser la question. Des filières industrielles, on a eu ce débat ces derniers ces dernières heures, on a eu ce débat sur la filière photovoltaïque, on a eu ce débat sur les éoliennes terrestres. Et aujourd'hui on a la chance de tenir sur la filière éolienne marine les briques d'une filière industrielle qui exporte qu'il a de l'emploi Net qui exportent aux États-Unis, qui exportent en n'Ecosse alors même que nous n'avons nous pas encore ou à peine commencé à installer des pales d'éoliennes des nacelles d'éoliennes, nous avons aujourd'hui les sites industriels qui fabriquent ces la bagatelle de 6500 emplois Directs à Cherbourg à Saint-Nazaire au Havre et effectivement, les élus sont inquiets par rapport à ces filières qui pourrait être fragilisée par le signal que nous allons envoyer en disant fabriqué chez nous, mais nous ne prendrons pas les fabrications que vous faites pour nos propres Park parce que nous estimons qu'il faut attendre d'avoir d'autres technologies il faut attendre de les mettre à 40 kilomètres de nos côtes, je pense que ce n'est pas tenable, sincèrement, je pense que ce n'est pas tenable au-delà de ça, je veux aussi dire une chose. L'article 12 telle qu'il est rédigé, il fait peser un très lourd contentieux sur les projets qui sont partis. Très lourd contentieux alors c'est pas les porteurs de projets qui vont avoir ce contentieux, c'est l'État qui aura défini les zones d'accueil des fameuses éoliennes ça va bloquer les extensions ça va bloquer des projets qui sont pas encore totalement attribué. Et puis moi je sais pas lire l'article qui dit évidemment on peut rerentrer dans les 40 kilomètres si il y a des raisons techniques, économiques qui font que, comment on l'apprécie ça. ça va être un nid à contentieux infernal. Donc je, je, à un moment où, justement, l'enjeu est d'accélérer notre production électrique, on sait que les éoliennes marines, c'est notre capacité à bâtir vite de fortes capacités de production, on sait que on sait pas aller aussi vite et aussi fort avec les éoliennes terrestres et avec le photovoltaïque, le photovoltaïque, c'est beaucoup d'espace et donc tout ce qu'on a fait aujourd'hui et que vous avez fait avec beaucoup de détermination, de trouver tous les espaces ou même des capacités de production électrique énergie d'énergies renouvelables, on reviendrait dessus avec cet amendement, je crois que ce n'est pas ce que nous voulons tous nous voulons tous de la production d'électricité bas-carbone nous voulons tous de l'indépendance énergétique, nous voulons tous de l'énergie à prix compétitifs, c'est ce que nous apporte ses installations et ce n'est pas tout à fait le même niveau de coûts pour des installations flottantes qui n'existe pas aujourd'hui, hein, je veux le dire aujourd'hui, au plan mondial, l'installation flottante, la plus aboutie, elle pèse 88 mégawatts. 88 mégawatts, pardon mais c'est rien du tout. Et donc nous sommes en train de mettre en danger une filière sur lequel aujourd'hui, nous sommes plutôt bon alors essayons. Peut être de ne pas reproduire ce que nous avons vécu sur le photovoltaïque, vous l'avez beaucoup évoqué cette perte de compétitivité, l'arrivée de panneaux. Venus de de l'étranger, en particulier de Chine aujourd'hui, nous avons dans nos mains la possibilité de construire une filière éolienne marine forte qui permettent de répondre à nos enjeux énergétiques, c'est pour cette raison que je demande la suppression de l'article 12. Ensuite, sur le 612 madame avait à la parole. L'article danser les alinéas 23 et 25 adopté en commission prévoit que les futurs appels d'offres, l'autorité administrative sélectionne des zones d'implantation située à plus de 40 kilomètres du Rivage, nous l'avons dit nous voterons contre, nous devons apprécier les projets au cas par cas dans un travail de concertation et de planification et on peut avoir un projet souhaitable à une distance inférieure et un projet qui ne l'est pas une distance supérieure en raison des activités en mer ou de l'environnement, pourquoi se priver a priori d'un tel espace ensuite avec une telle distance plancher d'implantation très éloigné de les côtes cela limiterait considérablement les zones éligibles et cette année ne euphémisme actuellement, à l'exception des parcs en centre Manche tous les parcs installés, de même que ceux en cours de développement sont à moins de 40 kilomètres des côtes alors reste le pari du développement de nos parcs éoliens sur les technologies flottante oui elle avance mais elle n'est pas encore mature, oui la France est le 1er pays à avoir lancé des appels d'offres pour des parcs commerciaux en Méditerranée et dans ma région, en Bretagne, mais il n'existe encore aucun parc commercial à ce stade, dans le monde, sans parler des postes de raccordement dans le pacte signé il y a quelques mois, l'État défend un déploiement ambitieux avec un objectif d'attribution de 40 Jiwa Gaouad installé en 2050 et j'ai rappelé aussi les engagements de la filière en introduction, il s'agit de soutenir une ambition forte et non de reculer. Nous poursuivons la discussion commune, nous avons encore six amendements donc nous examinons le quarante-quatre présenté par Messieurs Sautarel, vous avez la parole. C'est moi Monsieur Vial. Merci monsieur le président, mais mes chers collègues, on a bien vu qu'il y avait un petit malaise dans ce débat et que le seuil de 40 kilomètres qui qui faisait débat, alors là je vous proposer l'amendement de Monsieur Sautarel qui, qui vous propose de. d'apaiser ce débat en vous proposant un seuil à 25 les vingt-cinq mille nautique, ce qui représente environ 46,3 kilomètres mais, selon la formule qui peut le moins peut le plus, et donc, nous vous proposons cet amendement.

Oui, merci Monsieur le Président, donc c'est un amendement qui vise à permettre l'installation des éoliennes maritimes à une distance égale ou supérieure à 40 kilomètres de nos côtes, nous pensons que l'impact visuel est considérable pour avoir, en Loire-Atlantique Le 1er parc éolien Offshore au large du Croisic, je peux vous dire chers collègues, que le l'effet d'encerclement est saisissant et que vous les compter une par une, donc nous nous portons cet amendement à compter des prochains appels d'offres pour ne pas mettre en difficulté les appels d'offres déjà attribués. Si Monsieur saumon ensuite pour les 331. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi je trouve qu'on est assez loin de ce qu'on a discuté hier où on parlé de production par territoire et que l'Offshore paraît complètement indépendant

avec le nombre d'éoliennes que je vous ai cité déjà hier, si en plus on en est dans les Terres et qu'on nous en mais comme il est prévu en Baie de Somme ou à visibilité de la baie de Somme, vous voyez l'effet d'encerclement que nous pouvons avoir et la saturation que nous avons que nous quand on parle, qu'il y ait un partage, je dirais de l'effort territoriales,

d'existence déjà de de l'effort fait par les territoires et de l'effet d'encerclement ou de ou de dégradations, un petit peu du paysage et des zones touristiques que représente, en particulier la baie de Somme, donc moi je souhaiterais que, effectivement, de ce fait, on est plutôt favorable à avoir une distance qui soit supérieure à 40 ça pourrait être réduit si au moins deux fait on avait une étude d'impact qui tiennent en compte déjà de l'effort fait par les territoires et de l'impact visuel, que ça peut avoir aussi sur des zones touristiques dont on a dit tout à l'heure que le tourisme était une activité je crois très importantes en matière économique pour le territoire français. Monsieur Cabanel pour l'amendement 228. défendu tout à l'heure et qui, j'espère, tombera parce que je souhaite que se termine demain, comme tous les autres identique soient donc acceptées, il privilégie les zones d'implantation à moins de conflits d'usage lors des prochaines mise en concurrence des projets d'éoliennes en mer, a lieu et place de Ladislas minimale de 40 kilomètres des côtes. Et enfin, Madame Sylvie Robert pour l'amendement 532. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre amendement revient donc sur l'introduction de de cette distance minimale de 40 pour l'implantation des éoliennes en mer, en l'état cette distance apparaît totalement illusoire, aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue économique au regard des coûts de raccordement en d'autres termes, établir une telle distance signifie dans l'immédiat, freiner, freiner complètement le développement des projets éoliens en mer, voire au-delà de freiner concentrerait. Et je suis bretonne, donc je sais ce que en Bretagne dans les Pays de Loire, ces zones d'implantation, ce qui serait pas au demeurant complètement enfin étonnant mais surtout serait préjudiciable aux les fondements de la filière et donc à la protection des énergies renouvelables, mais ça reste quand même une dimension qu'il ne faut pas ignorer, à l'inverse, une distance de 12 milles nautiques, soit un peu plus de 22 kilomètres nous paraît être un juste compromis entre la foi, l'obligation de transformation écologique et des conditions plus réaliste d'ordre économique mais aussi technologique. Merci, alors nous allons passer l'avis de la commission, mais le président souhaite s'exprimer, vous avez la parole monsieur le président. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, compte tenu de la présentation des des amendements je vous sollicite pour une suspension de séance d'une dizaine de minutes. OK, donc nous disons que nous reprenons à 16

La séance est reprise. Donc nous allons commencer par l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements, discussions de séances mais le président Longeau demande la parole est là. Merci monsieur le président je je ne sais pas au niveau réglementaire, si ça se fait, mais j'ai demandé une suspension de séance, le temps est un tout petit peu court et ce qu'on peut avoir une nouvelle suspension de séance, en accord avec Madame la Ministre, pour terminer ce qu'on était en train de de faire et et et d'essayer d'écrire est-ce que ça vous va si on leur demande une suspension de séance, alors je je sais pas combien de temps ce que j'aurais pu dire les minutes le voulez après hein, on peut associer si vous voulez un représentant par groupe pour essayer de se trouver une solution. Non, Monsieur le Président, essayer de faire une évaluation tout de même que je puisse donner une heure de reprise. La ministre, ils me disent : trente trente minutes 30 minutes. ça compromet sérieusement la possibilité de terminer cette nuit. Donc, nous reprenons à 17 heures 20. Ou un peu plus tôt s'il y a un signal positif. La séance est suspendue.

La séance est reprise. Je donne à nouveau la parole au président Longeau qui va nous informer si je peux. Vous demander de reprendre votre place en séance, mes chers collègues, le président Longeau va nous exposer comment il voit la suite du travail. Avec un micro, ça serait mieux. Merci, merci bien, on va reprendre le cours de la séance, on a fait une une interruption de séance, mais on va examiner les amendements un par un, comme il était prévu et puis ma foi on votera, c'est pour l'instant, ce qui est ressorti de ski effectivement la négociation qu'on a eue avec. La ministre et les 5 membres de de commission.

la proposition que nous serions prêts à faire, c'est de partir de l'amendement de la sénatrice avait de le sous-amender au niveau du gouvernement pour permettre de nettoyer les sujets de distance, de manière à pouvoir voter derrière les amendements de suppression ou pas qui s'enchaînent, puisque si nous votions l'amendement de Madame avait on aurait un problème de faire tomber tous les amendements de suppression, je ne crois pas que ce soit le souhait sur ces bancs, et donc c'est la proposition que je vous fais, on va vous soumettre un sous-amendement.

de la commission sur le 622 dans son état actuel puisqu'il faudra le faire de toute façon. Oui, donc, la Commission avait un avis défavorable sur l'amendement 622.

On peut maintenir la séance si vraiment c'est une affaire de seconde pour établir un sous-amendement, mais il faudra ensuite que. Nous puissions a donné lecture.

Madame avait. Je crois qu'un sujet action. Qui paraît la plus expédiant c'est vrai que vous rectifiez votre amendement conformément à la suggestion qui est fait par les collaborateurs de Madame la Ministre, la rectification s'écrivait ainsi. Pour ceux qui veulent avoir le texte sous les yeux. Nous ne changerons bien sûr le grand hein et le grand de de l'amendement.

Je peux maintenant demander la ville du rapporteur sur l'amendement ainsi rectifié. C'est un avis de sagesse. Bien. L'avis du gouvernement. C'est un avis favorable, dès lors qu'il a été et permet le vote des amendements suivants. Ah. Oui, l'objet en effet de cette rectification et de ne pas. J'essaie de me faire comprendre l'objet de cette rectification et de trancher les points qui sont dans les trois premiers alinéas de l'amendement et de ne pas du fait de la discussion commune, faire tomber les autres amendements donc le Sénat se prononcera sur les amendements qui sont aujourd'hui prévues donc sous réserve de cette explication, je vous donne la parole, mon cher collègue. Oui j'ai peur de ne pas avoir tout compris. Donc, j'aurai besoin de d'éclaircissements sur ce que vous nous avez présenté est-ce qu'il est fait mention de la suppression de toute distance. réponse. J'essaie de comprendre. Non, non, non, Monsieur Gueï demande également la parole avant que la ministre précise l'explication.

comme je vois que personne n'a réussi à se mettre d'accord avec personne, bon il y a quand même des amendements de suppression. à mon avis, c'est plus simple de passer à ces votes là et après, de voir si on peut, bon, vous nous proposez un amendement rectifié mais personne ne comprend rien, je suis désolé, et c'est pas par manque de clarté, ni le gouvernement ni lui rapporteur ni de Monsieur le Président, mais en même temps, moins quatre, moins cinq, on retire, voilà la question centrale qui est politique, c'est ce qu'on reste au 40 kilomètres ou pas et c'est ça le débat. Et, bon ben après il y a des accords, des désaccords, vous avez compris qu'on est en désaccord avec ça parce que ça ne tient pas, d'un point de vue économique ça tient pas sur le raccordement bon bref, donc il faut qu'on nous explique politiquement

Il a adopté ou pas, mais il fera tomber les autres si on se mettent d'accord sur un amendement rectifier, je vois pas pourquoi après on irait supprimé l'ensemble des articles, donc voilà ça, plus rien, enfin ça a plus rien à voir avec ce que nous avions déposé dans les conditions dans lesquelles nous les avons déposé au moment où le le texte a été écrit par la Commission, donc, politiquement, il faut se mettent d'accord qu'est-ce que ça change, sur les 40 kilomètres une fois que nous avons tous compris, tout le monde vote en son âme et conscience et après on avance. Alors d'abord Madame avait et ensuite, Madame la Ministre. Alors, en fait, la rectification qui est proposé, c'est de ne plus faire référence à la ZE pour éviter que ça fasse tomber en fait systématiquement les amendements qui suivent. en fait ça ne ferait pas tomber les amendements de suppression derrière et on votera les amendements de suppression. La ministre. monde s'écoutent. Voter dans l'ordre les amendements tels qu'il se présente dans le déroulé de la séance, le premier amendement et l'amendement qui revient sur la rédaction. Ailleurs, en matière de et qui permet d'avoir des document stratégique de façade qui de permettent de concilier à la fois le dialogue public sur les éoliennes, mais de d'intégrer dans cette ce document stratégique de façade, les autres usages, les pêcheurs, les enjeux touristiques et etc. ça, c'est la correction apportée par l'amendement de Madame

ce qui est proposé. C'est d'enlever cette référence à une distance qui faisait tomber les amendements de suppression derrière sur lequel vous êtes plusieurs à vous être positionné de façon à ce qu'on puisse mener ce débat jusqu'au bout, soit les amendements de suppression sont et

discussion sur la discussion avec les les quatre amendements de suppression. Merci monsieur le président, moi je veux aussi repositionné sur le plan politique, les le, le débat qui est le nôtre actuellement et du coup éclaircir peut être la la position de la commission Culture puisque nous sommes un peu à l'origine, pas les seuls, mais de l'amendement des 40 kilomètres nous notre préoccupation est de ne pas refaire avec l'éolien maritime, ce qui a été fait avec l'éolien terrestre et ne pas provoquer les mêmes réactions de rejet sur l'éolien maritime qu'il y a aujourd'hui sur l'éolien terrestre alors peut être la tombe mal écrit à travers une question de distance pour lequel il n'y a pas manifestement de consensus mais néanmoins la préoccupation de dire ne refaisons pas les mêmes erreurs sur l'éolien maritime qu'on a fait sur les intéresse, elle reste présente à mon esprit, je, je reconnais que dans l'amendement de Madame il y a, il y a des avancées dans le domaine mais néanmoins je ne retrouve pas entièrement la préoccupation notamment par rapport au compromis, sur lequel nous sommes parvenus hier sur l'éolien terrestre à, à savoir le le le l'implication et le la concertation et les outils donner aux élus et aux conseils municipaux pour être pas pleinement partie prenante et puis aussi l'intégration de la problématique paysagère qui doit être prise en compte et qui n'apparaît pas en tant que telle, à ce stade, donc il y a une avancée à travers l'amendement, mais pour moi il n'est pas totalement satisfaisant. Il reprend la parole. Pour clarifier non. bien Monsieur Dantec. Madame Prima, demande la parole : ouais. Merci, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le rapporteur je je comprends pas bien en fait, ce qui est en train de se passer, pardon je je comprends que dans l'amendement de Madame avait on supprime donc la référence des 40 kilomètres

moi je me pose la question de savoir, on pourrait avoir un débat si vous preniez dans l'amendement de Madame avait c'est le souhaitait de rectifier cet amendement en faisant référence aux aider à Z E on pourrait avoir une discussion. juste une seconde, on pourrait avoir une discussion sur l'amendement de Madame avec qui comprendrait les et et qui anticiperaient entre guillemets sur une suppression parce que j'imagine que les nos collègues qui ont déposé des amendements de suppression peut être qu'avec cet amendement modifié qui n'a plus les 40 kilomètres mais qui a référence aux zones économiques ils enlèverai leur amendement enfin je fais peut être de leur amendement de suppression je je fais cette proposition parce que je pense que on pourrait trouver un chemin peut être, me semble-t-il. très très mal. Le rapporteur avant. J'avais demandé la parole depuis quelques instants, déjà je vais revenir tout de suite sur la vie que j'ai donné tout à l'heure qu'il est un avis de sagesse. L'amendement que nous avions proposé, qui a été adopté par la commission qui étaient intégrés dans texte était un amendement de compromis. Entre les mesures stricte d'éloignement des 40 kilomètres, on avait prévu quelque chose d'intermédiaire qui donnait la possibilité. Dans un certain nombre de situations après un ciblage prioritaire de pouvoir malgré tout venir en en deçà de cette limite. La discussion que nous avons eu tout à l'heure, je l'ai eue parce que j'ai vu l'amendement de Nadège avait et je lui ai demandé si on pouvait bâtir une proposition en commun sur la base de cet amendement qui intégré comme vient de l'évoquer, Sophie Primas la zone économique exclusive, et moi je me suis basé sur cette mention dans l'amendement pour donner mon accord dans la mesure où. Hou la mention n'y figure plus, moi, je donne un avis défavorable à cet amendement. Madame la ministre. pardon, je vais vous lire parce que, comme vous l'avez compris : on supprime le trois le le pardon, le 4 le 5 et le 6 mai il y a quand même une mention à la zone économique exclusive qui est dans le grand pour l'élaboration de la cartographie au 1er Rania du présent de sont ciblés en priorité des zones propices situé dans la zone économique exclusive donc qu'est ce que fait cet amendement, il dit que, de manière prioritaire va plutôt chercher à mettre des éoliennes marines dans la zone économique exclusive, mais ça ne l'impose pas. Et ça permet d'avoir la discussion sur la fin du texte qui impose une distance et donc à ce titre, il me semble, hein, et pour répondre à, à madame la présidente de la commission des affaires économiques, qu'on marque bien l'attention, l'intention de mettre au maximum des installations éoliennes marines au-delà de la zone économique exclusive, mais qu'on n'en fait pas un point d'accroche de contentieux en 10 ans. On s'impose de le faire au-delà, et si, sauf si il y a des soucis technologique et caetera, qui était le nid à ennuis qu'on avait repéré collectivement et par ailleurs, ça permet ou pas, d'avoir ce débat sur les 40 kilomètres qui est quand même un débat important, il y a des gens qui soutiennent les 40 kilomètres il y en a d'autres qui ne me soutiennent pas, il me semble que c'est porte de sortie, en tout cas, qui permet d'avoir ce débat démocratique. Monsieur Houlgate. C'est vrai que c'est un peu confus, moi personnellement dans dans les suppressions des Halles des alinéas, je ne vois pas la suppression de l'alinéa 23 qui fait justement référence à la distance minimale de 40

le le de la distance à 25 milles nautiques, je propose au rapporteur ou à Madame la ministre, de faire un sous-amendement Mandement puisqu'ils sont les seuls à pouvoir le faire et de simplement sous-amendé, c'est de cet amendement Sautarel pour remplacer 25 milles nautiques par 25 kilomètres

et qui pourrait peut-être satisfaire la plupart d'entre nous. Je rappelle que nous avons 11 amendements en discussion commune. Et que donc le Sénat ne pourra se prononcer que lorsque l'avis de la commission et du gouvernement aura été sur les 11 s'il y a la possibilité. Qu'un amendement simplifie la discussion et il me semble que nous n'y sommes pas. Et je donne la parole au président Karoutchi mais je crois deviner sa pensée. Je vais éviter de me prononcer sur l'éolien maritime mais en revanche, monsieur le Président, Madame la Ministre, lorsque, il y a suspension de séance pendant finalement près d'une heure, soit il y a un accord global. Sur la modification de l'amendement, soit il y a pas et s'il n'y a pas, on reprend le cours normal du débat pour être plus clair et chacun s'exprime comme il veut, parce que pardon de vous dire que depuis une heure, on n'y comprend plus rien, plus personne ne sait où sont ses petits moi je propose que Madame avait conserve son amendement d'origine qui a un débat et puis chacun vote en conscience sur l'ensemble des amendements qui ont été déposées, parce que là franchement arriver à quelque chose qui n'a pas de sens, au bout d'une heure pour dire que de toute façon qu'on parle même pas de ce qu'on va voter non, on fait une modification en séance si y a un accord entre la Commission, le gouvernement, les groupes et on avance, mais si c'est pour n'arriver à rien, restons-en au débat classique normale. Je crois que ça ne pourrait être le cas. Au terme d'une nouvelle suspension dont je ne suis pas sûr qu'elle soit fructueuse. Donc j'ai donné la parole à la ministre, mais sur le plan de la méthode, il me semble que c'est le président Karoutchi qui a raison et qu'il faut bien que nous passions au vote complet si si Madame avait même. Tiens, la modification de son amendement on le votera modifiée mais on le votera après examen de tous les autres, donc Madame la Ministre. Non, mais j'ai Houlgate, pardon mais. ce ne amendement que nous avions déposé, c'était tout simplement au niveau de l'alinéa 23 remplissait les 40 kilomètres par les 12 milles nautiques, ce qui fait un peu plus de, de, de 22 kilomètres peut constituer le sous-amendement de l'amendement rectifié de Madame avait.

on peut décider de faire remonter le vote sur l'amendement de suppression, sur les 40 kilomètres, c'est-à-dire le 227 336 584 et 612 et après ceci étant nettoyer l'amendement de Madame avait prend tout son sens et c'est la discussion qui est dans le bon sens, il me semble, il me semble, moi, c'est la proposition que je vous. Simplement, simplement la règle d'examen du texte, si je peux arriver à me faire entendre. La règle d'examen du texte et qu'on ne peut. Examiner les amendements en discussion commune, c'est-à-dire ceux qui s'excluent mutuellement que ensemble, donc la solution. Me paraître que le rapporteur exprime l'opinion de la commission et le Gouvernement ensuite sur les 11 amendement en sachant qu'ils sont exclusifs les uns des autres et qu'ensuite nous réserve sur la demande du gouvernement ou de la commission, le vote des 2 premiers amendements pour statuer en premier sur les amendements de suppression. Qui sont en discussion commune. Monsieur le rapporteur, veuillez donner l'avis de la commission de façon méthodique, s'il vous plaît, sur les 11 amendement dans l'ordre. ça va être très mais méthodique, monsieur le Président, je dirais même presque chirurgicale puisque c'est un avis défavorable sur chacun des amendements. Madame la ministre. C'est un avis favorable sur les amendements six cents. 227 336 584 et 612. Et défavorable sur tous les autres. Je vous je vous consultez sur 11 amendements.

Nous allons donc nous prononcer si le gouvernement demande la réserve des votes madame la Ministre. Est ce que vous demandez la réserve des votes sur les 2 premiers amendements. Donc nous allons voter et sur la base un scrutin public sur les amendements de suppression qui porte le numéro 227. 336. Voilà quoi. La commission et le groupe LR nous ont fait parvenir une demande de scrutin public. Mes chers collègues, le groupe LR maintient-t-il sa demande de scrutin public.

le groupe LR maintient sa demande de scrutin public. Bien sûr. Donc nous avons un scrutin public. Sur cette série de 4 amendement 227 336 584. Et 612 qui sont identiques et qui supprime les amendements 23 et 25. Le scrutin est ouvert.

Je répète, personne ne demande plus à voter. Le scrutin est clos. Les résultats du scrutin votants 340 exprimés 337 pour les amendements 186 contre 151 donc les amendements de suppression des alinéas 23 et 25 sont adoptés. Dans ces conditions, nous reprenons la suite. Des amendements réservé sachant que le vote de ces amendements de suppression fait tomber les amendements, si je peux avoir votre attention 199 331 228 et 532 reste donc à soumettre au vote du Sénat, le premier amendement le 622 de Madame

Si la dope la demande de scrutin public sur cet amendement est maintenu ou non. Non, donc nous allons procéder pas à main levée sur le vote de l'amendement de Madame avait rectifié. Qui est pour. Non, c'est une rectification. Donc, qui est pour l'amendement de Madame avait rectifié. Un invité sur la radio. Qui a un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement. Oui, j'ai bien dit défavorable de la commission. Bon, qui est pour cet amendement.

l'amendement 447 de monsieur Lahellec qui n'était pas en discussion commune et donc soumis à une discussion maintenant et monsieur Lahellec le présente. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement 447 : nous l'avions envisagé. Pourquoi. Dans l'hypothèse où nous n'aurions pas commis les votes qui viennent de se dérouler autrement dit cet amendement visait un objectif. D'avoir de l'ambition pour l'implantation d'éoliennes, y compris dans l'hypothèse où. Les 40 kilomètres nous aurait été imposé. ça n'est pas le cas, nous tenons compte des scrutins précédents et par conséquent nous nous proposons de retirer cet amendement. C'est logique monsieur le mon cher collègue, et donc on ne se prononcera pas sur cet amendement, qui est retiré. Nous pensons ensuite sur au vote sur la Lire l'article 12 ainsi. Il y a pas de demande d'explications de vote, donc je le soumet au vote du Sénat qui est pour l'article 12. Qui est contre. Il est adopté.

pour essayer de rattraper le temps il est défendu. Je ferai de même défendu. Monsieur le rapporteur, avis défavorable sur ces deux amendements, madame la ministre. Avis favorable aux voix ces deux amendements de suppression du 12 bis avec un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement, quels sont ceux qui sont pour.

Après l'article 12 bis, nous avons un amendement 310 de Monsieur Dantec. merci monsieur le le président, hein, donc, cet amendement vise à expliciter la possibilité qu'à l'état d'attribuer les lots à plusieurs opérateurs de manière à démultiplier les retombées industrielles et limiter les risques de non-réalisation des objectifs de développement de l'éolien en mer personne en situation de de monopole. Je mets aux voix cet amendement 310 avec un double avis défavorable qui est pour. Contre. N'est pas adopté, je mets donc aux voix, l'article 12 ter nouveau.

Contre. Il est adopté.

elles sont continuent à des mères territoriales dans l'activité économique, pêche, tourisme, sport et aussi la réimplantation des coraux sont de la compétence régionale ou départementale et quelquefois même communal parce que ça se fait à Saint-François pour les coraux notamment, il semble donc légitime de permettre aux collectivités territoriales, qui sont à proximité de ces zones d'émettre un avis sur les autorisations d'exploitation d'énergies maritime sur ces zones frontalières, je vous remercie. Quel est l'avis de la commission monsieur juste un avis défavorable. Madame le ministre, oui, l'amendement est satisfait et donc demande de retrait.

ça paraît logique, monsieur le rapporteur, un peu plus de précisions. D'accord avec Madame la Ministre, alors nous ne sommes pas défavorables au fait de consulter les territoires ultramarins préalablement la délivrance d'autorisation d'implantation pour les parcs éoliens dans leur zone économique exclusive, cependant, cet amendement est satisfait : l'article 13 ne modifie pas les modalités d'association des territoires ultramarins aux décisions d'implantation d'installation dans leur zone économique exclusive, c'est donc le droit commun en matière de consultation des collectivités d'outre-mer qui s'appliquera donc il est pleinement satisfait. C'est également votre avis, Madame la Ministre. Donc il est satisfait et vous le retirer, nous pouvons donc nous prononcer sur l'article 13 qui est pour l'article 13. Contre. Il est adopté. L'article 13 bis ai l'objet d'un amendement de précision qui est présenté par monsieur le rapporteur, le 656. Le président, un amendement de précision rédactionnelle. Le ministre Je mets aux voix cet cet article avec cet cet amendement proposé par la Commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Contre et il est adopté, et l'article 13 bis, hein. Modifié même vote. Il est adopté, je mets aux voix, l'article 13 nouveau qui est pour. Contre. Abstention : il n'a pas, il est adopté à l'article 14 de nouveau un amendement de la commission 657 monsieur le rapporteur. En correction : l'Égypte. Madame le Ministre.

pour. Il est adopté, et l'article 14 qui est pour. Contre. Il est adopté à l'article 15 est un amendement qui tombe. Et donc je mets aux voix, l'article 15 qui est pour. Contre. Il est adopté, après l'article 15. Nous avons un amendement de monsieur Calvet et de ses collègues, il est défendu par Monsieur Moga, qui a la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le présenteras 22 vise à accélérer le traitement des dossiers d'instruction et de délivrance des projets pour l'éolien en mer aujourd'hui, les délais d'instruction et de délivrance des autorisations sont de 12 à 15 mois l'objectif de réduire à neuf mois ce délai a été énoncée par le conseil général de l'environnement et du développement durable dans le cadre de son rapport sur la simplification des procédures d'autorisation applicable aux éoliennes en mer, publié fin 21 l'accélération des délais d'instruction des dossiers se fait sans préjudice du reste du respect des exigences environnementales et des règles de procédure. Amendements identiques de monsieur Montaugé qui a la parole est à monsieur le président, il est défendu, c'est strictement la même. L'avis de la commission monsieur rapporteur. Ces amendements sont pleinement satisfait par l'article 1er que nous avons voté et nous avons introduit par ailleurs les amants les article IV bis pour accélérer la phase d'autorisation administrative des projets, c'est donc un un, un avis défavorable, parce que ça. Madame le Ministre : avis défavorable également. Donc ces amendements sont, d'après le rapporteur satisfaits sont-ils maintenus.

Nous avons un amendement de suppression et présenté par Madame pareil pour peut être finalement les trop vite de choses sont surprenantes dans cet article : la première serait de vouloir faire travailler des entreprises pas encore désignée lauréate en leur confiant la rédaction d'une convention pour laquelle il n'est pas encore officiellement prévu que l'entreprise soit payé la 2ème chose surprenante, serait de savoir à l'avance qui va emporter une procédure de mise en concurrence, marché avant que le jury ne se soit prononcé dans les 2 cas, il y a un problème de transparence et de déontologie et donc un problème de philosophie de l'action publique, les chantiers engendrés par le développement des énergies renouvelables, son tout comme leur montant et nous ne pouvons pas les confier en acceptant une opacité ouvrant droit à des dérives, nous proposons donc de ne pas statuer sauter les étapes et de ne pas anticiper la décision d'un processus de désignation qui doit demeurer souverain. favorable, monsieur le président. Madame la ministre. C'est un avis favorable votre amendement vise à supprimer l'article 15 bis qui prévoit que l'État signe la convention d'occupation pour l'éolien en mer avant le résultat final de l'appel d'offres, le gouvernement rappelle qu'il était défavorable à l'introduction par la commission de cet article 15 bis, car cette mesure conduit à délivrer la concession d'utilisation du domaine public maritime très en amont, sans avoir connaissance de l'étude d'impact du projet et sans consultations préalables tels que l'enquête publique, cette mesure nous semble contraire au principe constitutionnel de non régression protégé par l'article 1er de la charte de l'environnement, toutefois, le gouvernement ne partage pas l'année Anne-Lise selon laquelle le fait d'avoir conclu la convention là. La CUD PM influencerait le choix du lauréat final pour le coup, puisque le lauréat final sera le même que lauréat pressenti, désigné par le ministre en charge de l'énergie, sauf s'il est dans l'incapacité de répondre à ces obligations, constitution des garanties, notamment si un nouveau lauréat pressenti devait être désigné, alors c'est à lui que serait attribué la concession, quoi qu'il en soit, j'émets un avis favorable sur cet amendement. Je consulte le Sénat sur cet amendement 437 donc un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour.

Il est adopté. Et du coup, l'article est supprimé. à l'article 15 terre nous avons de nouveau un amendement de numéro 448 présenté par Monsieur là, elle qui a la parole. nous souhaitons réaffirmer la priorité à la concertation et à la prise en compte des exigences formulées par les collectivités, qui devrait, à nos yeux primer sur l'article 15 terre évidemment l'article 15 terre nous paraît complètement indispensable pour définir une stratégie nationale, mais l'objet de cet amendement vise à permettre à ces collectivités d'être réellement entendu dans le cadre des procédures merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, je partage évidemment l'esprit de cet amendement, sensible aux aux énergies marines renouvelables, l'article ne concerne que la planification des implantations installations de production d'énergie renouvelable terrestre et non les énergies marines renouvelables qui sont visés par l'article 15 Des actions et investissements en faveur de l'adaptation des infrastructures portuaires au développement des derniers des énergies marines renouvelables c'est une compte des choix qui seront actés par les acteurs locaux en matière d'implantation de parcs éoliens en mer comme prévu à l'article 12 je pense cependant qu'Achoui qu'ajouter cette précision dans la loi n'est pas indispensable, c'est donc un avis défaveur. Madame la ministre. Sur le 440 8 un avis également défavorable.

Nous votons sur l'article 15 ter cher collègue qui est pour. Qui est contre. Il est adopté Nous avons un amendement 620 de Madame avait. L'amendement vise à rétablir la rédaction initiale. Monsieur le rapporteur, vous pouvez donner l'avis de la commission sur cet amendement 620 s'il vous plaît. Merci monsieur le le président le rétablissement, l'de l'article 16 initial n'est pas souhaitable car il reviendrait à supprimer le cadrage institué par la Commission en 1er lieu à la souhaité cibler les ouvrages de raccordement sur ce électrique de plus à la entendu confier la compétence au représentant de l'État dans le département et prévoir la consultation de la commune ou du groupement de communes et, le cas échéant de la commission départementale de protection des espaces naturels, la autre point : la commission a souhaité privilégier l'enfouissement des ouvrages sauf dérogation environnementale enfin la exclu ces ouvrage volumineux du décompte de l'objectif 0 artificialisation nette Lausanne ces garde-fous sont légitimes dans ces c'est dans ce cadre que je fais une demande de retrait, sinon ce sera un avis défavorable. Qui est l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Votre amendement vise à rétablir l'article 16 dans sa rédaction initiale, j'y suis favorable toutefois, je vous propose de codifier l'Arctique qui supporte les dispositions concernées en mentionnant qu'il s'agit de l'article L 121 5 2 du code de l'urbanisme je ai j'aimais donc un avis favorable sous réserve de cet ajustement de forme. Madame avait d'accord avec la suggestion de la Ministre sur le l'inscription donc la la l'inclusion dans le code, s'il n'y a pas d'autres interventions je soumets au Sénat cet amendement 620 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission est d'un avis favorable du gouvernement qui est pour.

oui, donc la la la la, l'amendement de 620 réécrit l'ensemble de l'Arctique, il fait donc tomber l'ensemble des autres amendements touchant à l'article 16 qui est ainsi rédigé et qui est donc voté. Avant le 16 bis, nous avons à l'amendement 450 qui est présenté par Monsieur Gremillet. merci, monsieur le président, madame Nice, monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement prévoit tout simplement qu'un décret en Conseil d'État détermine les critères selon lequel le renouvellement d'un parc éolien doit ou non être regardés comme constituant une modification substantielle par rapport au code de l'environnement, un incident et l'obtention d'une nouvelle autorisation environnementale.

Je demande la sagesse du Sénat sur cet amendement. Madame la Ministre. Votre amendement propose de préciser par un décret en Conseil d'État, les critères. Permettant de considérer le renouvellement d'un parc éolien comme substantielle ou non cette appréciation qui relève d'une Ali d'une analyse au cas par cas par l'inspection de l'environnement, s'appuie sur un cadre qui est déjà défini au niveau de circulaires les critères à considérer pour définir si un nouveau si un renouvellement de parc éolien terrestre et notable substantiels sont déterminés dans l'instruction du gouvernement du 11 juillet 2018 relatives à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres cette instruction établit les critères et seuils d'appréciation permettant de juger du caractère substantiel de la modification qui décide de la nécessité d'une nouvelle autorisation ou non je tiens toutefois vous assurer qu'un travail approfondi est en cours pour préciser ses. Critères pour les inspecteurs, parce que je pense que c'est aussi à l'attention de de votre part, en préservant le principe selon lequel toute création de nouveau donne lieu à une nouvelle demande d'autorisation et en clarifiant les règles applicables oripeaux je dirais que d'une certaine manière votre amendement est satisfait puisque le travail est déjà en cours, pas forcément au même niveau de réglementaire, mais pour la souplesse, la rapidité, c'est une demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur Daumier. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre. Oui. Merci pour la vie du de notre rapporteur de sagesse effectivement. C'est je, je, nous savons tous ce qu'il a déjà quelque chose qui existe, sauf que, entre ce qui existe et ce qu'on vient de faire, il y a d'autres éléments a intégré. Madame le Ministre je vais vous faire confiance, vous vous engagez effectivement à modifier, à intégrer effectivement ces nouveaux éléments, à partir de ce moment-là, je considère qu'effectivement il est satisfait. Donc je le retire. C'est logique, donc, nous passons aux amendements sur l'article 16 bis et nous avons 2 amendements. Identique qui réécrivent l'article qui seront donc vote pour l'article en même temps, donc c'est d'abord l'amendement 599 du gouvernement et le 629 ensuite de Madame avec. Oui, madame, mais en premier, si le gouvernement préfère. Vous donnez votre appréciation sur l'amendement avait surtout vous défendez le vôtre. Donc l'amendement du gouvernement mais je crois qu'il est dans le dérouleur oui. Il vise à revenir là l'amendement qui qui a été adopté en commission. sur avis favorable sous réserve du gouvernement avait pour objet de prévoir la prise en charge de radars de compensation pour les installations de la Défense, il serait intéressant d'étendre cette disposition également au radar de la navigation aérienne civile et aux radars de compensation pour météo France, donc c'est ça qu'il s'agisse de s'appuyer sur la rédaction du de la commission et de l'élargir à 2 autres objets dans le même esprit de faciliter les l'installation d'énergies renouvelables. Nous avons donc et 2 amendements identiques qui réécrivent l'Arctique et qui font l'objet d'un avis favorable de la commission qui est pour. L'abstention, ils sont adoptés et donc l'article 16 éteint 16 bis est ainsi rédigé après le bis, nous avons un amendement 526 ce qui est présenté par Monsieur cardons et qui est défendu par le même Merci monsieur le président je vais, je vous propose de présenter l'amendement 526 et l'amendement 535 en même temps pour l'amendement 526 le présent amendement propose d'instaurer une garde au sol minimale de passage de la pale à 30 mètres pour les parcs éoliens cette disposition entend ainsi indiqué le phénomène de surmortalité des oiseaux et des des chauves-souris aujourd'hui qui est constaté au pied des éoliennes présentant un quart de sol de moins de 30 mètres pour l'amendement 535 les parcs, les projets de parcs éoliens ont l'obligation légale de déposer à la Caisse des dépôts et consignations, une somme proportionnelle à la puissance des machines pour permettre leur démantèlement complet, néanmoins il apparaît que certains démantèlement ont engendré des coûts bien plus important que les sommes cosigné. Ah. Pardon, ce risque est par ailleurs d'autant plus grands dans un contexte inflationniste et cet amendement propose donc la création d'une commission indépendante présidée par un membre de la Cour des comptes qui serait chargée d'étudier le caractère approprié des garanties financières apportées et l'opportunité de réévaluer à la hausse les montants qu'ont consigné. Il s'agit d'un enjeu crucial pour notre territoire, il faut éviter que les parcs éoliens d'aujourd'hui ne deviennent les friches de demain, je vous remercie.

la garde au sol et cetera, c'est donc un un avis défavorable. Madame la Ministre avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement de Monsieur carton numéro 526 avec un double avis défavorable qui est pour.

Après le seize bis toujours j'ai un amendement 200 du président va et de ses collègues, il est défendu par Monsieur de Nicolas qui a la parole. Oui, monsieur le président, le présent amendement vise pour les installations produisant de l'éolien à faire de la conciliation entre les mains de la Caisse dépôts et consignation la modalité unique de constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état des sites après exploitation, ce dispositif vise à sécuriser les porteurs de projets, les sommes consignant consigné étant protégé, sécurisé rémunéré tout au long de l'exploitation des parcs éoliens, il permet également de renforcer l'acceptabilité des projets auprès des riverains, les fonds nécessaires au démantèlement étant déposée auprès d'un tiers de confiance opérant en toute neutralité. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur, un avis favorable à cet excellent amendement. Madame la Ministre. envie de pouvoir assurer ses opérations en cas de défaillance les dispositions relatives aux garanties financières ont été renforcés en décembre 2021 donc désormais aux 50000 euros précédemment applicable s'ajoute un montant supplémentaire de 25000 euros par tranche de 1 mégawatt au-delà de 2 mégawatts pour la puissance de la machine ainsi les éoliennes plus puissante et plus grande sont soumises à des obligations supérieur et donc il me semble que votre amendement est satisfait pour précision à ce stade, mais il ne faut pas préjuger de l'avenir, il n'a jamais été nécessaire de faire appel à ces garanties supérieures financière c'est pourquoi je, je, c'est une demande de retrait. Madame Lavarde demande la parole. pour autant, que se passe-t-il quand les entreprises qui ont exploité ont fait défaut. Et qui enfin comment est pris la garantie, c'est un peu ce que sous-tend en fait ces amendements de c'est quand on est l'entreprise qui a construit qui, pour laquelle la garantie n'est plus là, on se trouve avec des corps morts qui sont toujours sous terre, donc l'objectif en fait était de s'assurer que les sommes consignées dans le cadre où là, dans le cas où l'entreprise ne perdurerait pas pourrait bien être appelé au moment où il s'agit de démanteler les installations si on ne fait pas de reporting.

qu'on le garde pour l'autre loi sur le nucléaire et qu'on propose, qu'il a un tiers de confiance qui, effectivement, l'ensemble des sommes de déconstruction de toutes les installations de production d'électricité, je pense qu'il y a une idée là qu'on va approfondir. Après cet instant de créativité, ce qu'il y a d'autres interventions, Madame la Ministre. En fait, donc si je comprends bien la un amendement l'idée de dire le tiers de confiance et la Caisse des dépôts par rapport à des banques qui assure ce service, sauf qu'aujourd'hui, les banques sont bien dans une prestation, on n'a jamais eu de difficultés avec ses banques d'abord donc, sauf à ce que vous ayez un cas mais ou un précédent et par ailleurs il y a un problème conventionnel qui est lié au fait que ces banques proposant ce service qui est une prestation de marcher, il paraît difficile de leur confier le monopole à la Caisse des Dépôts, donc voilà mais. Donc. Nous avons cet amendement avec un avis favorable de la commission. Défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Et il est adopté. Nous revenons à l'amendement 535 messieurs Cardon a soutenu tout à l'heure, il porte également sur les sujets de. Consignation, l'avis de la commission. Et défavorable et là. La ministre également défavorable. Je me vois cet amendement 535 de monsieur qui est pour. Qui est contre. si je peux avoir l'attention des collègues. Je crois qu'il est adopté.

Le vote a eu lieu, nous avons ensuite un amendement de Madame Lherbier dans télé seul signataire et je ne la vois pas. Ensuite, nous avons un amendement dont le premier signataire et monsieur Bachere.

l'excavation systématique de l'atelier de de la totalité, parlons des fondations des éoliennes jusqu'à la base de leurs semelles, est un gage d'acceptabilité locale des projets pour les riverains des parcs éoliens et les communes sur le territoire desquels sont situés ses projets cet amendement garantit également une remise en état optimal du terrain compatible avec l'exercice des activités agricoles. Monsieur le rapporteur qu'est l'avis de la commission. C'est un avis défavorable, cet amendement est satisfait par l'arrêté du 22 juin 2020, je vous invite évidemment à consulter avec la plus grande attention. son auteur, le retire, enfin un de ses auteurs, le retire monsieur Cardo ensuite. Merci monsieur le président, cet amendement donc 534 sur le balisage lumineux le balisage lumineux fait régulièrement partie des griefs opposé au parc éolien, notamment la nuit, période durant laquelle ses effets sont encore plus ressentie par la population, limiter le balisage lumineux, c'est limité le les potentiels nuisances ressenties fin 2021 une expérimentation a été initiée pour diminuer le balisage lumineux dirigée vers le sol et ne laisser que celui vers le ciel, une autre expérimentation a été lancé en Ardèche pour étudier les possibilités de déclencher le balisage nocturne uniquement au passage des dans la mesure où les résultats de ce expérimentation n'ont pas été transmis au Parlement, cet amendement impose au gouvernement de produire un rapport exhaustif sur les expérimentations réalisées et de le remettre au Parlement, je vous remercie. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. et d'identifier les pistes d'évolution en la matière, plus sérieusement, c'est une contrainte et nuisances souvent cité, donc c'est un avis favorable. Madame la Ministre sagesse. Donc l'amendement de Messieurs cardons. Et soumis au vote avec un avis favorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Bon contre. Il est donc adopté.

ce présent amendement vise à réintroduire une annexe sur la situation hydroélectriques existantes dans le bassin au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le stage.

Après l'article 16 toujours, nous avons six amendements identiques, le 1er est celui de Madame Goulet. Et certains de ses collègues Madame Deckers le le Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, cet article donc présenté par et Madame Boulay, mais aussi Madame Billon Calvé vise à augmenter le potentiel de développement de la petite hydroélectricité sur des moulins hydrauliques existants pour l'essentiel est estimé au minimum à 290 cependant la remise en eau et la remise en service de ces s'ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde souvent incompatibles avec l'importance technique et économique de l'ouvrage qui bride considérablement et qui rend impossible la mise en oeuvre de tels projets, il s'agit donc d'un article additionnel afin de de lever les obstacles réglementaires liées à la remise des services de ses ouvrages afin de produire de la petite. aucun des signataires de l'amendement n'était présent, et donc il est tombé. Le vingt-huit rectifié de monsieur de Nicolas et de ses collègues, c'est pour ça que je suis présent. Bien

Monsieur le Président, Madame la Ministre, le développement du du développement, la petite hydroélectricité sur les moulins hydrauliques existants pour l'essentiel est estimé comme l'a dit ma ma collègue qui n'avait pas le droit d'en parler, mais qui en a parlé quand même depuis plusieurs années, toutefois, alors même que la plupart de ses ouvrages sont fondées en titre autorisé au code de du code de l'énergie, comme du code de l'environnement et qu'en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisés rapidement l'administration a multiplié les obstacles et c'est vrai réglementaires liées à leur comportement, leur remise en haut et leur remise en service, en exigeant moultes prescription dissuasive et onéreuse, je dois dire que cet amendement a été c'était signé par un très grand nombre de, de, de collègues qui prouve combien les élus sont attachés à la présence des Moulins et de la petite et et de électricité sur notre territoire.

est qui est appelé ou qui devrait être appelée à à se développer encore, notamment par rapport à la petite rideaux hydraulique, donc la proposition de céder cet amendement elle est très simple : il s'agit, concernant le confortement la remise anneaux et la remise en service et d'installations qui ont été autorisés, ancienne avant le 16 octobre 1919 pour une puissance modeste n'excédant pas 150 qui kW/h de ne pas être de n'être soumis à aucune formalité autre qu'une information du du préfet comportant, le cas échéant et limitativement l'identité du du propriétaire, et le quasi-et de l'exploitant, ainsi que la localisation précise l'installation de l'ouvrage ou des activités, donc c'est une simplification administrative qui irait dans le dans le redonner une une seconde jeunesse à des à des installations très anciennes qui pourrait tout à fait être remise en service. Toujours dans ces amendements identiques chez Monsieur, Corbizet ce qui défend le 114. Je pas quand même dans la ami comme mon collègue mais Riou a copié mon amendement est défendu. Ensuite, le 100 89 et défendu par Madame Saint-Pé. Vous êtes signataire, ma chère collègue, vous le défendez, il est défendu et enfin, et nous avons Madame Ract-Madoux. Donc, quelle est la ville de la commission sur ces six amendements qui sont identiques. Le président nous avions souhaité dès l'origine, je l'avais évoqué d'ailleurs dans la discussion générale, hier matin, introduire l'ensemble des énergies renouvelables dans ce texte, donc avant de vous donner la vie, sur ces six amendements, je voudrais simplement préciser que sur les sur certains des suivants, il y aura des avis défavorables des avis favorables, pardon, mais c'est un avis défavorable sur ces six amendements. Madame le Ministre. Avis défavorable également. Bien. Eh bien nous, monsieur Montaugé. merci Monsieur le Président, bon d'accord j'ai j'ai on prend acte de la position de la Commission et du gouvernement mais je on on aimerait avoir quand même quelques arguments à l'appui de cette position de refus catégorique, merci d'avance. lui vaut mieux que vous avez priorité. 1919 sans autre formule alité qu'une déclaration et sans possibilité pour l'État diffère opposition or depuis la loi de 1898. C'est bien 1800 hein, la mise en place d'ouvrages sur les cours d'eau et soumise à autorisation de l'État et les autorisations sont équivalentes à des autorisations environnementales à condition d'être toujours subsistent tente, ainsi, l'État doit contrôler d'abord si l'autorisation antérieure et subsistance et doit pouvoir s'opposer à la mise en service d'ouvrages qui ne dispose plus de titres et deuxièmement si les modalités de remise en service d'un ouvrage qui dispose d'un titre permettent le respect des objectifs issue du stage, comme toute autre autorisation environnementale et le cas échéant, doit pouvoir imposer des équipements permettant d'assurer cette compatibilité pour le dire en des termes plus clairs, là on va tellement à la simplicité qu'en fait on remettrait en état des ouvrages qui sont très anciens, sans réellement savoir si c'est compatible avec notre droit de l'environnement, donc il me semble qu'il faut le retirer, j'émets un avis défavorable sur cet amendement. Avant 2020, monsieur le président, le ministre des membres de la commission aménagement du territoire, nous avons été reçus au Conseil d'État et a été évoquée lors de discussions, la problématique des Moulins, or les Moulins, c'est presque un Dora séculaire, c'est-à-dire que pas du moment où vous à un moulin qui est inscrit dans la carte de Cassini, le propriétaire d'un moulin aujourd'hui est en droit de produire son électricité, il faut déposer un permis demande d'autorisation, mais le préfet, les services de État ne peuvent pas s'y opposer, c'est-à-dire que tous les recours en haut tribunal administratif au même au Conseil d'État, les propriétaires ont eu gain de cause, donc ça remonte bien plus loin que 1800 et des brouettes, donc je crois qu'à un moment donné, moi je ne veux pas qu'on cède au lobby des pêcheurs parce qu'aujourd'hui on a déjà eu un débat ici ou les lobbies des pêcheurs aujourd'hui or sont tellement puissants, que dans les agences de l'eau, on donne maintenant des subventions pour détruire les Moulins alors qu'il y a quelques années, on en est, pour les remettre en état, c'est pas pour autant que les propriétaires des moulins ne sont pas dans l'obligation de remettre des passes à poissons ça Fillon c'est autre chose, effectivement, là, dans le cas des thèmes on ne serait dans l'obligation dans de mettre une passe à poissons, pour que les poissons remontent, mais en tout cas, ça reste un droit séculaire et tous les candidats au recours ont tous gagné l'Euro Oui, je crois que il est assez évident qu'on ne peut pas repartir comme ça avec des autorisations aussi ancienne notre rapporteur a peut-être été un peu laconique sur le fait de savoir quels amendements il allait soutenir, il me semble notamment que tout le travail qui a été fait en commission du développement durable pour justement trouver un compromis sur cette question et qui avait été fait par Pascal Martin était un bon équilibre, donc est-ce qu'il y aura un soutien à l'amendement Martin enfin c'est important qu'on sache vers quelle amendement de compromis et en fait de dialogue, on va, si c'est celui, Pascale Martin je pense qu'effectivement, ça serait une bonne solution

mais vous les avez vus en commission, enfin pour ceux qui sont de la commission, en tout cas, donc j'y reviendrai tout à l'heure, alors après leur présentation. Monsieur Folliot, vous demandez la parole. merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'hydroélectricité, la première, énergies renouvelables, d'un autre pays. Et, et, depuis quelques années, je veux dire, non seulement de tous les grands projets sont arrêtés mais aussi tous les petits projets qu'il peut y avoir ici ou là par l'inflation ne normes administratives que nous avons mis en place donc sont complètement bloqués, moi je partage tout à fait les propos que vient de tenir notre collègue parce qu'ils sont empreintes de bon sens de logique et cet amendement est un amendement qui va dans le sens de somme toute non pas Madame la Ministre, de créer de nouvelles infrastructures simplement de rap remplacer des installations hydroélectriques très vieillissante par de nouvelles, moi j'ai un exemple dans mon département, la commune de Mirandole Bourguignat qu'elle hein, une petite centrale hydroélectrique très vieillissante avec du matériel qui date d'il y a dire dire très longtemps et pour le remplacer, oh, on lui demande des autorisations à n'en plus finir, on lui demande de faire des aménagements qui peut pas ça, poissons et autres alors que cette chaussée, elle existe depuis des siècles et des siècles, nous ne sommes pas dans des schémas qui sont des schémas raisonnable je crois que cet amendement va dans un cadre non pas de simplification, mais du Biarritz du bon sens, comme on dit chez nous et et je crois que ça me paraît important de les soutenir et de les voter, parce que cela va faciliter le développement de petites installations hydroélectriques qui contribueront à cet objectif majeur que nous avons de promouvoir les énergies renouvelables Merci monsieur le président, madame la ministre, nous le savons tous aujourd'hui, il y a recul très important de la biodiversité et les signaux sont de plus en plus alarmant aujourd'hui sur ces reculs, or en terme de biodiversité dans le milieu aquatique, un des facteurs qui est déterminant, c'est la rupture des continuités écologiques qui fait qu'aujourd'hui, notamment les poissons migrateurs mais l'ensemble des poissons qui qui vont frayer ne peuvent pas remonter les cours d'eau et les frayères comme ça devrait être normal et donc on a un niveau de reproduction qui est particulièrement faible dont tout obstacle aujourd'hui aux continuités écologiques participent à l'effondrement de la biodiversité, ça c'est le 1er point et le constat général qui est indéniable, le 2ème constat c'est que l'ensemble de ces politiques de l'eau, au moins sur 90 % ou 80 % se situe aujourd'hui dans des stages. Dans des sages dans des programmes d'action accepter, négocier politiquement avec des syndicats de rivières, des EPAGE, des EPTB sur lesquels ce programme d'action participe de la reconquête de la continuité écologique, revenir sur ses principes, c'est remettre en question également la délibération collective, tout le processus d'élaboration autour de ces documents de plan d'action et de mise en oeuvre de l'ensemble de ses programmes avec les financements associés au niveau des comités de bassin, donc on peut très bien entendre le respect patrimonial, mais ne tient pas, par ailleurs en terme d'impact cette petite hydroélectricité ne pèse que 0 5 ou 1 % à l'échelle nationale et est très relative aura au regard des enjeux de développement des énergies renouvelables.

j'ai pas l'impression que le problème de la continuité écologique a été gêné depuis depuis le XIVe siècle, non, ce que ce que je veux dire sur cet amendement, c'est, c'est très simple, je crois que notre collègue corriger l'a très bien expliqué on peut faire de la petite hydroélectricité ça ne gêne pas la seule chose que demande ce qui sont propriétaires de moulins c'est que puisqu'ils sont fondés en titre et qui gagneront

de toute façon ils vont gagner et ce qu'il demande simplement, c'est qu'on leur fasse on aurait on reconnaisse une fois puisqu'ils vont gagner en reconnaît cela et que ils puissent accélérer et faciliter la mise en place d'une petite hydroélectricité c'est simplement alors si on veut supprimer les l'hydroélectricité sur les petites rivières et les barrages, ça c'est une autre politique, je comprends ce que veut dire gilet en disant les barrages ne sert plus à rien mais bonjour moi je, enfin nous avons-nous sur le Loir, pour prendre un exemple, beaucoup de barrages, les agriculteurs sont extrêmement sensibles à cause des problèmes de d'irrigation à la présence de barrages et Les Halles petite hydroélectricité permet là aussi de, de, d'avoir un rôle dans la dans la dans la transition énergétique et, surtout, la production d'énergie. Je voudrais dire 2 mots seulement sur le dogme qui ait porté actuellement qui consiste à prétendre que, aujourd'hui, l'existence des Moulins et contraire à la bonne tenue de la biodiversité, c'est une, c'est une erreur fondamentale, il y a 100 ans, 200 ans, il y avait des poissons partout donc aller chercher ailleurs, si vous voulez, les raisons de la dégradation des eaux et de la biodiversité, ce sont probablement des problèmes de pollution qui n'ont rien à voir avec les moulins, donc je pense que ce dogme doit être revu. Oui, monsieur le président, je ne vais pas rajouter beaucoup de ce qui vient d'être dit à l'instant. Mais sincèrement. Quand vous êtes sur le terrain. On a tous. Quelques cheveux blancs. Et donc, on a quelques années derrière nous. Et pourquoi j'évoque cela, je vais l'illustrer je vais confessé à cet instant que je suis un pêcheur de vendre dans tous les sens du terme. Et dans mon petit village, mais c'est du concret. Dans mon petit village et un petit ruisseau qui s'appelle la bouillante qui passe devant moi mon exploitation qui prend sa source à même pas un kilomètre. Il y avait. Quatre Moulin une fécule un tissage et j'ai toujours attraper détruite en dessous au-dessus, j'ai toujours pêcher des écrevisses en dessous et au-dessus, donc ce qui a été fait par nos ancêtre, on vient de pas de nulle part. On doit être capable de continuer le préserver et n'oubliez pas que la France, on parlait tout à l'heure du bilan carbone, on parlait de de produire nos panneaux photovoltaïques en France mais n'oubliez pas que la France est le 1er pays à travers le monde. Qui a le la capacité de produire des turbines. Et là encore, comme aujourd'hui, tout est à l'arrêt tous les progrès qu'on aurait pu faire sur l'amélioration la productivité de la production électrique de ces turbines dans ses petits moulins, même si c'est pas grand chose, moi on m'a toujours appris hein et hein ça fait deux et ce qui est petit et grand parce que lorsqu'on assiette un additionne les petites choses, ça représente beaucoup pour nos territoires. Et quand je vois tout à l'heure. Ce qu'on a été capable de faire, à juste titre sur la préservation de notre Patrimoine. Mais là aussi, c'est toute l'histoire de notre pays, on a une richesse dans nos départements, dans nos territoires de cours d'eau qui ont été capable de produire de l'énergie, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on serait plus capable d'en produire. Monsieur mais de vielle qui a demandé la parole qui là. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je pense que tout est question d'équilibre, moi je vais aussi d'une vallée où le le seul sport praticable, été la pêche à la main, on peut le dire, maintenant il y a prescription, j'étais assez sportif mais à à l'époque il y avait des des populations de je pense aux migrateurs à l'anguille saumon qui était supérieure de de 95 % oui nous avons perdu sur les 50 dernières années 95 % des populations, alors il y a aujourd'hui 5000 ouvrages sur les rivières françaises si avec si on avait gardé le même taux de population, évidemment, il y a d'autres facteurs, la disparition, il y a la pollution il y a eu les nitrates ça poserait pas de problème, mais là avec le le le niveau actuel de population, on va vers une disparition de ces espèces, si on ne se met pas, si on met pas aux normes, certains Moulins, je crois qu'il existe aujourd'hui des turbines horizontale qui permettent quand même de limiter les effets, c'est moulins, donc restons prudent quand même et surveillant la population parce que sinon, ça serait quand même un désastre d'avoir des rivières sans truites et sans écrevisses Daniel. Monsieur Vial.

même si je comprends qu'il peut y avoir des des enjeux réglementaires, il y a un dogme que mon mon collègue Favreau a voulu démonter tout à l'heure, je partage absolument son son avis moi je voudrais en démonter un autre quand on nous parle

qui fonctionne au chantage avec les élus locaux, en nous disant : vous, vous vous avez le droit à des subventions sur l'eau et sur l'assainissement, vous ne les aurez que si vous mettez en oeuvre le le l'arasement de tels seuil où de tels barrages ou d'hôtel Moulin c'est une forme de chantage, alors si vous appelez ça le consensus et la démocratie, je suis désolé, on est on pour moi, on est très au-delà de de ce que j'appelle, moi, la démocratie, donc, ça remet pas en cause les enjeux et les intérêts des uns et des autres mais mais de grâce ne, ne nous dites pas que c'est la volonté partagée de l'ensemble des élus de fonctionner de cette manière, c'est : on n'a pas vraiment le choix. Le Sénat me semble suffisamment éclairé, donc je vais mettre aux voix, les 6 amendements identiques. Quels sont ceux qui sont pour. Alors. quels sont ceux qui sont contre. Donc ils sont adoptés. Après l'article, Esther, nous avons un amendement. De monsieur Pascal Martin de 311 qui est défendue par le président Lo'Jo. Merci monsieur le président, mamie, ces travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, on on revient à ce sujet parce que. Je vais qu'on évoquait tout à l'heure, avait déjà été évoquée dans la loi qui a été voté au mois d'août l'année dernière c'était le rapport de Guillaume Chevrollier, qui était rompre avec la continuité écologique destructive réconcilier préservation de l'environnement, activités humaines ont montré que la mise en oeuvre du principe de continuité écologique

que des incompréhensions subsistent toujours et que le dialogue entre l'administration et les propriétaires de moulins à eau demeure difficile dans certains territoires, la mise en oeuvre d'une politique de continuité écologique apaisée et réellement une nécessité la libre circulation des espèces aquatiques et le bon transport des sédiments permettent d'atteindre l'objectif de bon état écologique des masses d'eau fixé par la directive-cadre sur l'eau de 2000, il est tout autant nécessaire de tenir compte du potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques et la valeur patrimoniale des moulins à eau une solution équilibrée et de bon sens pas, ce n'est certainement pas la réconciliation des acteurs chargés de la restauration et du maintien de la continuité écologique, c'est la raison pour laquelle le présent amendement institut une médiation en cas de désaccord entre l'administration et un propriétaire d'ouvrages, plutôt que de je dis judiciariser la procédure, source de lenteurs et génératrice de frais de justice pour les propriétaires, il est proposé d'instaurer une solution reposant sur la médiation par l'intermédiaire d'un référent territorial désigné, désigné par le préfet, cette mesure est proposée dans le but de favoriser le développement du potentiel de la petite hydroélectricité, c'est cette solution est d'autant plus que la sévérité de la sécheresse, était et a montré cette année que des conflits d'usage des ressources en eau était désormais possible dans notre pays à climat tempéré. l'avis de la commission. Oui, monsieur le président de l'instauration d'une procédure de conciliation en cas de désaccord sur les modalités de maintien de restauration de la continuité écologique est une bonne idée, je crois pas je fais bien les arguments de du président et c'est donc un avis favorable. La vie de la ministre. La loi climat et résilience a prévu que les porteurs de projets ou les gestionnaires d'installations hydrauliques pouvait solliciter une conciliation amiable en cas de désaccord, cette disposition a été intégrée dans l'article L 220 ans 14 17 1 du code de l'environnement, cette même loi prévu la mise en place d'une expérimentation de médiation un médiateur des enjeux de préservation de la continuité écologique et de développement hydroélectrique a été désigné en Occitanie, pour une durée de 4 ans, et donc c'est une proposition de retrait ou avis défavorable. Monsieur Corbizet. Madame la Ministre, cette médiation, elle existe en Occitanie dans d'autres départements, il y a pas de conciliateur et si on compte sur la DDTM pour être conciliateur, ça veut dire que c'est même pas la peine de présenter un projet Eole, expliquez moi j'habite à côté d'Arras, ma maison, coincé entre le canal de lascars avec une écluse et l'autre côté, ah, dernier bras de la rivière ce carte après un moulin donc dit : tiens,

dit au moins de ça d'être entraînée par Sergueï Boubka je ne vois pas comment ils vont faire un bond de 3 mètres mais je dis l'autre côté de ma maison, j'ai une écluse qui souffrent de 3 fois par semaine, donc vos poissons, il y a pas de raison qu'il passe pas par l'écluse, bon,

Et ce qu'il y a d'autres explications de vote monsieur Favreau. Ce qui est proposé, nous connaissons bien la façon dont, actuellement, les syndicats de rivières sont tenus par les techniciens de rivière qui reçoivent les consignes directement. Du ministère de l'environnement et des agences de l'eau et nous savons très bien comment finalement aujourd'hui tous les moulins sont attaqués sur nos rivières de France, c'est parce que, effectivement, il n'y a pas d'égalité dans la discussion lorsqu'on évoque les sujets techniques qui permettent de restaurer la qualité des eaux puisque vous avez d'un côté, des techniciens qui sont formés, instruits par le dogme que j'évoquais tout à l'heure et les gens du terrain, les riverains qui sont tenus à l'écart de toutes les dispositions qui sont prises. Moi je trouve que c'est une excellente proposition que d'instaurer de façon visible et quasi systématique puisque ce sera instauré un lieu de médiation qui va au moins sur les moulins dans un 1er temps mais peut-être nous servir dans d'autres cas pour trouver le juste équilibre entre les différents usagers exigence de l'eau, je le dis d'autant plus que j'ai été la rapport triste au Parlement européen, donc celle qui a négocié au nom du Parlement européen la directive-cadre sur l'eau et nous avons eu de longues discussions sur justement le risque qu'il avait de trop normé autant l'exigence bon état écologique définition du bon état écologique était devait être très rigoureux autant la manière d'y parvenir devait autant que faire se peut développer des lieux de consensus ou en tout cas de de rendre lisible les enjeux et d'arbitrage et dans cet état d'esprit, moi je considère que la France, notamment quand on a dû ratifier par la loi sur l'eau n'a pas beaucoup développé dans la mise en oeuvre de la directive, tout ce qui était conciliation concertation implication des différents acteurs, je l'avais regretté à l'époque j'avais des regretter notre tard aussi, je pense que les agences de l'eau non non pas non plus beaucoup agi avec en étant proactif, je rappelle que, on est encore avec plein de territoire qui n'a pas atteint les objectifs de la directive qu'on devait déjà avoir atteint et donc, il me paraît en tout cas important que ces cultures de la médiation sur le bon usage de l'eau évidemment dans le respect des règles du bon état écologique se développe dans notre pays. Monsieur Gillet reprend la parole. pour essayer de proposer des médiations intelligentes qui permettent, le cas échéant de maintenir des seuils, mais à partir du moment on a aussi des solutions de continuité écologique, il faut essayer de négocier avec les parties prenantes donc sur le fond, c'est une voix effectivement médiane qui peut être intéressant mais pour répondre quand même ah monsieur Favreau sur les syndicats de rivière, d'abord ils sont présidées par des élus, et c'est eux qui embauchent, donc ils ont quand même la responsabilité de l'employeur et même les syndicats de riz, les techniciens sont quand même sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle des responsables, des élus qui siègent au niveau des syndicats de rivière et sur les syndicats de rivière, l'ensemble des parties prenantes sont associés les plans d'action sont validés de manière collective, donc si on veut vraiment poser des sujets il y a un lieu de débat pour pouvoir le faire.

Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement donc déposé par monsieur Gremillet, Rémy Pointereau et de nombreux collègues vise à lever les freins au développement de la petite hydroélectricité en précisant que les services instructeurs des demandes de remise en exploitation d'ouvrages potentiel hydroélectrique veillent à ne pas faire peser sur les propriétaires ou les gestionnaires des 10 ouvrages des charges qui obèrent équilibre financier de leur projet à cette fin, le présent amendement précise à l'article L 214 17 du code de l'environnement que les prescriptions émanant des services de l'État en matière de continuité écologique intègre la nécessité de ne pas pénaliser l'équilibre financier des projets en tenant compte de la disproportion qui peut exister entre certaines mesures de franchissement demander et les capacités financières des propriétaires ou des exploitants, il est en effet important de soutenir la petite hydroélectricité une énergie décarbonée.

sauf que là on parle de des usines qui ont dispensé qui seront dispensés d'autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance consistance légal déterminé en appliquant la même formule que celle qui figure au 3ème alinéa, c'est-à-dire que ce qui nous permet, effectivement, là encore, de rendre possible l'exploitation dans ces périmètres dits de la petite Hydro-sur nos territoires. La visite de la commission sur ces deux amendements, monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Ces. Vise à ce que les services de l'État en matière de recommandations sur le fondement de la politique de continuité écologique veillent à ne pas pénaliser l'équilibre financier des projets, donc ce qui est plutôt louables et vertueux, donc c'est un avis favorable sur ces deux amendements. Sur les deux Madame la Ministre, ces 2 avis défavorable, défavorable, Thierry de. Je mets aux voix d'abord l'amendement 413. Avec un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour.

la loi d'énergie et climat de 2019 acté l'urgence écologique et climatique, il a rappelé spécifiquement dans le code de l'énergie, la nécessité d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, cette loi est insuffisamment suivies d'effet car les schémas de planification sur l'eau, les agisse d'âge prévu dans le code de l'environnement et pas dans le code de l'énergie, non pas de mission explicite d'intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydroélectrique ce nouvel article rend explicite et opposable fait que les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau et des et des territoires garantissent désormais la participation de l'énergie hydroélectrique à la décarbonation du mix énergétique français. Et un autre amendement émanant de d'autres collègues du groupe de l'Union centriste et du RDSE, dont Madame Saint-Pé est présente. Merci monsieur le Président, dames, la ministre de la Langlois énergie qui mettent de 2019 acté l'urgence écologique et climatique et a rappelé spécifiquement dans le code de l'énergie, la nécessité d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, cette loi est insuffisamment suivies d'effet car les schémas de planification sur l'eau prévue dans le code dans de l'environnement et pas dans le code de l'énergie, non pas de mission explicite d'intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydroélectrique, il en a résulté de dommageable mesure dans la décennie 2010 encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombres d'ouvrages producteur d'énergie hydroélectrique ou pouvant l'être facilement ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau et des territoires garantissent désormais la participation de l'énergie hydroélectrique à la décarbonation du mix énergétique énergétique français, il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d'un ouvrage peut être rétabli de multiples façons compatible avec l'exploitation énergétique. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces trois amendements. C'est un avis défavorable sur ces trois amendements. Et le 4ème amendement en discussion commune. Madou dans ces dans ses signataires, donc vous avez la parole, ma chère collègue. Il vient d'être défendu par ma collègue Saint-Pé. C'est pas tout à fait le même, mais si il est défendu, il est défendu la la vie du de la commission sur le 373, monsieur le rapporteur, un avis défavorable. Défavorable. Oui. Madame la Ministre, sur ces quatre amendements défavorables sur les quatre. Donc je mets aux voix d'abord les trois amendements identiques, enfin les deux qui reste parce que, hein, il tomber, donc les 30 et 191 qui ont fait l'objet d'un avis. Défavorable à chaque fois de la Commission et du gouvernement qui est pour. pour. Ils ne sont pas adoptés. Oui. Et l'amendement 373 monsieur Lou et de ses collègues, avec le même double avis défavorable qui est pour. Compte. Il n'est pas adopté non plus toujours après le secrétaire nous avons. Une nouvelle série d'amendements identiques portant article additionnel nous commençons par monsieur

régulièrement installés sur les cours d'eau inscrits en liste de à cette fin, il complète l'article L 214 tiré 18 du code de l'environnement, en précisant que ce régime d'exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique afin d'assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l'eau ainsi que du règlement anguilles.

était présenté pour partie par mon collègue Jean de Nicolas il est je compléterai en indiquant que cet amendement veillent également aux bonnes relations entre les services administratifs et les propriétaires ou gestionnaires des moulins à eau en instaurant une obligation pour l'administration de motiver les prescriptions complémentaires de gestion, d'entretien et d'équipement des Moulins, au regard des engagements européens, je vous remercie. qui a jugé l'article L 214 tiré 18 tirer hein contraire aux engagements européens de la France parce que le régime d'exemption des règles de continuité écologique pour les Moulins où était incompatible avec les objectifs de la directive cadre sur l'eau et le règlement anguille, nous ne parlons pas de le présent amendement précise par conséquent que les services de l'État peuvent prescrire des mesures de franchissement des espèces piscicoles, en dépit du régime d'exception d'exemption fixées par le législateur en 2017, l'administration est en revanche tenu de motiver ses demandes complémentaires au regard des engagements européens, donc un avis favorable sur ces deux amendements Madame le Ministre. Cet amendement vise à faire perdurer l'exonération. Sont des obligations au titre de la continuité écologique pour les cours d'eau, classé en liste de que le Conseil d'État vient de déclarer non conforme aux obligations européennes, L 214 18 introduit une exception par rapport à l'article L 214 17 qui impose de regarder au cas par cas les impacts des ouvrages situés sur 11 pour 100 des cours d'eau métropolitain où l'enjeu de continuité écologique a été jugé prioritaire le Conseil d'État, par décision du 28 juillet 2022, a constaté l'un conventionnel IT de l'article L 214 18 hein qui exonérer tous les moulins des obligations d'équipements permettant d'assurer le respect des obligations de continuité écologique ainsi le Conseil d'État a estimé que les ouvrages ne peuvent pas être exonérée des obligations d'équipements pour la continuité écologique, de manière générale, le premier alinéa de votre amendement revient à appliquer ce qui est déjà prévue prévue par l'article L 214 17 donc a priori il n'est pas utile, il est également contraire au sens de l'arrêt du Conseil d'État qui avait reporte sur l'État, la charge de la preuve de l'impact de l'ouvrage sur le milieu et créent une rupture d'égalité injustifiées vis-à-vis de toute autre ouvrage que des moulins ayant les mêmes caractéristiques physiques vis-à-vis de centrales hydroélectriques plus puissante qui se situerait sur le même cours d'eau, or la puissance espérée de ces moulins n'a rien d'équivalent, c'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur votre amendement. C'est un problème constitutionnel oui. Je mets aux voix ces amendements avec un avis favorable du rapporteur de la commission et un avis défavorable de la près de la ministre. Qui est pour.

Ils sont adoptés après l'article Esther. Dans six amendements en discussion commune nous commençons par deux amendements identiques, du moins. S'ils S'ils ont des signataires présents le 1er ce n'est pas le cas. Le second si Madame P. et Monsieur saumon sont présents. Donc, le 193. Demande de madame Loyer, président alors que le développement de la petite hydraulique reconnu comme étant d'intérêt général que le contexte de crise énergétique actuelle rend plus nécessaire que jamais, la mobilisation de ce potentiel locale et décentralisée, il est dès lors proposer de le vers les freins réglementaires introduits au cours des dernières années et de consacré par la loi, les principes dégagés par le Conseil d'État en matière de définition de la puissance au consistance légale donne droit fondé en titre et d'une autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique, délivré avant 1919.

Oui merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, je propose de présenter le trente-cinq et le trente-six et puisqu'ils sont similaires, c'est-à-dire de c'est le calcul de détermination de la puissance par rapport à la consistance légal attaché à un moulin est déterminée par la formule qui figure au 3ème alinéa, donc c'est par rapport au calcul de la chute qui détermine, calcul de la puissance. Sur ces amendements, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. La, la, la commission souhaite garantir et préserver le régime d'autorisation, donc, c'est donc un avis défavorable sur chacun de ses 6 enfants. Avis défavorable. Alors je commence par l'amendement six qui reste. Non, c'est le contraire : c'est le 193 qui reste autant pour moi. donc avec un double avis défavorable, quels sont ceux qui sont pour.

L'amendement 374 qui a été défendu. Même vote aussi. Et les amendements présentés par Monsieur Gremillet, je commence par les 35 qui est pour.

C'est le 516. Monsieur Gillet. là sa squatter introduit en commission vise à permettre à l'autorité administrative en cas de tensions sur le système électrique de pouvoir fixer des débits minimaux temporaire inférieurs à ceux prévus actuellement par la loi, actuellement, l'article 214 tiré 18 du code de l'environnement précise que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit permet de maintenir dans celui-ci ah début minimales garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les zoos au moment de l'installation de l'ouvrage, il précise également que ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du Module du cours d'eau en aval immédiat ou aux droits de l'ouvrage correspondant des mi-moyens intérêts annuels cet article prévoit déjà la possibilité de fixer des valeurs de débit minimal selon les périodes de l'année dans des cas précis, les auteurs de cet amendement donc s'inquiète à l'heure de la multiplication des crises : énergétique, économique et climatique que nous traversons et des aléas qui les accompagnent que des situations de tension sur le système électrique soit amené à se multiplier dans les années à venir, et par là même que les dérogations fleurissent, il rappelle que la rédaction actuelle de l'article vise simplement à permettre que la vie demeure dans nos cours d'eau, ce qui semble être un objectif prioritaire, il semble en conséquence très inopportun de permettre une telle dérogation à l'heure où la France ne respecte toujours pas ses engagements européens ont beau en matière de bon état écologique de ces cours d'eau, en outre, nous interrogeons sur le réel impact d'une telle dérogation pour les ouvrages de la production hydroélectrique qui pourraient être concernés par cet article lors d'une période de crise ou des tensions qui le justifie, c'est pourquoi elles estiment également fortement précité de permettre une telle dérogation en l'absence d'étude d'impact.

il ne s'agit pas d'un dispositif et une idée inédit, pardon, puisque l'article L 214 18 du code de l'environnement prévoit déjà que des débits inférieurs puisse être fixés par elle, selon la période d'étiage, naturellement, il ne s'agit que d'une faculté et non d'une obligation de plus, nous avons prévu que ce dispositif ne puisse être appliquée qu'en cas de tension et qu'à titre temporaire, restons-en au texte issu de la commission, c'est une demande de retrait sinon défavorable. C'est un avis favorable parce que la faculté pour le prix. Fait de fixer des des des débits inférieurs au débit minimum à mentir pour les cours d'eau en cas de tension sur les réseaux, ça existe déjà, vous le savez, pour des motifs d'intérêt majeur et pas seulement en cas de tension sur le réseau électrique, et donc je pense qu'il faut trouver ce juste équilibre pour des motifs évidemment d'intérêt majeur, c'est-à-dire réellement une très forte tension et on a pris des dérogations, on peut le faire, j'ai pris des dérogations cet été alors la cité relatifs à la température mais ça revient au même, en revanche, l'idée c'est de ne pas le faire à chaque fois qu'on a une tension générale aujourd'hui on pourrait dire on a des inquiétudes sur l'approvisionnement en électricité, on va changer les les étiages je ne pense pas que ce soit une bonne chose, il faut avoir ce juste équilibre entre et notamment pour maintenir le respect des engagements européens en matière de bon état écologique des masses d'eau, je rappelle que le le combat à venir, ça va quand même être la perte de dos, enfin en tout cas la la baisse de nos cours d'eau dans le cadre du réchauffement climatique et qu'on va vite avoir à à trouver des des points d'équilibre entre les différents usages de de ça et donc il faut être d'ores et déjà très vigilant à ne pas rentrer dans des conflits d'usage qui existent déjà et qui sont complexes.

Défavorable de la commission est favorable du gouvernement ah excusez-moi, nous avons une demande de scrutin public du groupe, les républicains et donc il va être procéder au scrutin public dans les conditions de l'article 56 du règlement.

Et donc, le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin votants 343 exprimés 343 pour 146 contre 197 donc, cet amendement. Pas adopté, nous passons.

je m'interroge, mais je le présente quand même le présent amendement vise à limiter la possibilité pour l'autorité compétente d'abaisser le débit minimum réservé des cours d'eau en cas de tension forte sur le système électrique ou sur l'approvisionnement en électricité à la seule période hivernale, le débit réservé permettant de maintenir la vie aquatique dans les cours d'eau, de respecter les droits des usagers situé en aval ne convient pas d'autoriser cette diminution aux périodes pendant lesquelles les conflits d'usage de l'eau pour les plus fortes. Merci monsieur le président, la mention de la période hivernale, proposé par l'amendement n'est pas utile d'une part, elle est assez flou et ne figure ni dans le code de l'environnement, ni dans le code de l'énergie, d'autre part, elle ne correspond pas nécessairement aux besoins enfin mon amendement 564 qui va vous proposer une rédaction meilleur de cette périodicité vous l'aurez dans quelques instants, dans l'attente, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame la Ministre.

le présent amendement a pour objet de fixer des conditions d'application entre entre l'article Cesc inquiet, c'est l'Arctique ces pièces en faisant ainsi référence à une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement, ainsi qu'à une période d'application. Et la présidente, qui va nous donner l'avis de la commission. Sur un amendement dont elle est co-signataire mais oui : avis favorable, oui, on pouvait le deviner, madame la Ministre défavorable. Donc nous avons l'amendement 564 avec Ali favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour.

Il est adopté.

Puisque c'est soit les débits minimaux. Soit, en réalité, l'augmentation de la puissance, donc c'est la même chose. Nous, nous proposons que ça soit sous l'autorité administrative parce que comme Madame la Ministre, l'dit : nous vivons un stress hydrique. Malheureusement, avec le la question du dérèglement climatique. Les conflits d'usage. Vont s'accélérer. Il y aura besoin à un moment donné. Notamment sur la question hydroélectriques soit à mon avis beaucoup plus de puissance, mais il faudra faire attention évidemment aux autres, notamment sur la question agricole et donc nous ne sommes pas contre. Le fait que nous ayons recours à des dérogations. Mais il faut strictement les encadrer en tout cas, qui a un regard de l'autorité administrative, donc le 400 mètres et le 421 plus tard, c'est la même défense d'amendements, je vous remercie. Le suivi environnemental proposé par l'amendement n'est pas nécessaire tout d'abord les diminutions de seuils sont déjà l'objet d'un tel, suivie de la part du gestionnaire de l'installation, comme de l'autorité administrative de plus le dispositif proposé par l'article 16 quater prévoit que les mesures ne puissent être prises qu'en cas de tension et qu'à titre facultatif et temporaire, c'est donc une demande de retrait ou d'Avis défavorable. La ville, le gouvernement Madame le Ministre, gouvernement. ça sera un avis de sagesse parce qu'à partir du moment où on a élargi les situations où on pouvait baisser les débits, il va falloir suivre la baisse de ses débits et pour le moment effectivement l'article L 214 18 prévoit un suivi mais que pour les motifs d'intérêt majeur et donc, il me semble qu'il faut adapter, par contre, en terme de rédaction je recommanderais qu'on puisse le regarder dans la navette. Donc nous avons sur cet amendement 420 un avis défavorable de la commission et un avis favorable, enfin ou de sagesse du gouvernement, interprété par interprété par monsieur gay et donc je le mets aux voix, quels sont ceux qui sont pour.

Contre il était adopté. Nous passons au c'est qui, inquiet sur lequel le président Gontard, a demandé la parole il là.

avait oublié la question de l'hydroélectricité et c'est vrai que quand on parle de d'ENR, sans parler d'Hydro-ça peut poser quand même question c'est quand même la première source d'électricité renouvelable en 2 % en France et donc je pense que c'était important qu'on puisse même évoqué cette cette problématique de l'hydro-et notamment du du gros Hydro-et des barrages de plus qu'4 5 gigawatts c'est vrai que cette disposition de l'article de l'article 16 avec ce principe de consignation proposés dans dans le texte et à la fois intéressantes mais ne règle pas tout et surtout pointe justement la question des concessions et des concessions qui sont arrêtés, qui sont et sur lequel on a cette incertitude puisque ben ces concessions n'étant pas renouvelé la question de l'investissement, la question de la sécurité, donc on voit que c'est une situation dans laquelle on ne pourra pas rester très longtemps on a proposé plusieurs solutions, notamment la question de la de la quasi-régie qui serait une solution 100 % public et une solution qui respecte le droit européen, il me semble qu'il s'agit d'un enjeu de souveraineté de de pilotage sur le réseau électrique et de gestion de l'eau et qui est un enjeu de plus en plus majeure du coup, les orientations en tout cas sur cette question là du du gouvernement et puis sur le, sur le développement d'Hydro-on sait que l'effort doit être mis aussi sur les stations de transfert d'énergie par contact par pompage hein les steppes qui est un un des dispositifs renforçant la pilote habilité du système électrique, et donc le développement des des nous proposions d'exonérer les nouvelles stations des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité pendant 10 ans, mais bon, l'Arctique 40 est passé par là et mais je pense qu'il y a une réflexion à conduire sur en tout cas l'exonération de l'IFER et puis la loi fixe un objectif de doublement des capacités de stockage d'électricité hydraulique d'ici 2030 et je voulais savoir ce que prévoit le gouvernement pour justement tenir cet objectif et développer les les Alors, si le premier amendement en discussion et, le 375 qui est présenté entre autres par Madame Ract-Madoux voilà, si vous avez la parole chers collègues. Monsieur le président, cet amendement vise à faciliter les investissements de maintien en très bonne état des concessions hydroélectriques comme on vient de l'évoquer en délais glissants, afin de ne pas dégrader la performance de ses installations jusqu'au renouvellement des concessions, il vise tout d'abord à préciser les investissements pouvait être inscrit sur les comptes dédiés pour éviter tout effet indésirable ou double comptage et il permettra aux concessionnaires de réaliser des investissements dans des concessions échues depuis parfois plus de 10 ans, il impose également avant toute demande d'inscription sur ce compte dédié d'établir l'état des dépendances de la concession sous la forme d'un procès-verbal contradictoires entre l'autorité administrative et le concessionnaire afin de garantir que les investissements inscrits sont éligibles à ce compte dédié.

il revient sur le travail de la commission d'autre part, il est contraignant, s'agissant de ses modalités d'application réglementaire, enfin je lui préférerais une rédaction plus plus souple, telle que celle proposée par l'amendement qui va suivent le numéro 412 c'est donc une demande de retrait ou sinon un avis défavorable.

Oui merci monsieur le président, n'a un ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, effectivement, cet amendement a pour but de d'apporter des précisions techniques du travail qui a été fait par la commission. L'avis du rapporteur de la commission. en août, elle permet de spécifier une procédure idoine, enfin, contrairement à l'amendement 375 que nous venons d'examiner, elle s'insère correctement dans le texte de la commission, c'est donc un avis favorable. Madame la ministre, je vous demande l'avis du Gouvernement sur l'amendement 412. alors si je comprends parfaitement l'objectif parce que, effectivement, je je le partage de la rédaction ne me semble pas correspondre tout à fait à cet objectif et donc c'est un avis défavorable. Messieurs Gremillet le maintenu. Sans commentaire, merci donc je mets aux voix cet amendement numéro 412 madame la présidente de la commission souhaite s'exprimer. Monsieur le président, très vite pour défendre finalement cet amendement donc j'entends le j'entends les les critiques qui sont émises par Madame la ministre, ou en tout cas les interrogations, donc moi je propose qu'on l'adopte et qu'on le travail pendant la la navette. Bien ça n'accélère pas le rythme mais ça clarifie le dialogue, donc je vais vous mettre. Oh voit donc cet amendement 412 avec un la vie maintenant favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Ah bah oui, qui est contre, ça a fait de l'effet donc. L'amendement 565 c'est monsieur Gagnier qui le présente aussi. Oui, monsieur le Président, ça est très rapide, c'est du rédactionnel précision rédactionnelle. Du la commission.

pour. Qui est contre. Il est adopté, nous nous en venons au vote sur l'article qui est pour l'article 16 qui acquiesce. Le vote pour l'article cher collègue qui est pour. Y a-t-il des contre, il est adopté après. Nous entrons dans l'article 16 sexy S et nous avons 2 amendements

ces comités sur la consulter sur les seules décisions à évaluation environnementale au lieu des décisions il un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, pour rappel, ces comités sont composés de représentants de l'État des établissements publics du concessionnaire des collectivités territoriales et le regroupement des riverains, mais aussi d'associations représentatives d'usagers de l'eau, alors que le réchauffement climatique provoque davantage de tensions en matière de gestion de l'eau, l'ajout de cette mesure ne semble pas pertinent, la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique adopté ici en 2021 proposé d'accroître la formation du comité de suivi sur toute évolution dans l'organisation des installations hydrauliques, nous comprenons mal pourquoi on viendrait dans ce projet de loi réduire ses compétences. Monsieur Montaugé pour le l'amendement 543 identique. Oui, monsieur le président merci à maman identique, on n'est pas pour la restriction des des compétences et du périmètre cette commission importante. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, les amendements 258 et 543 sont identiques, il propose de supprimer l'article 16 sceptique issu des travaux de notre commission, la commission a souhaité moderniser le fonctionnement des comités de suivi de l'exécution des concessions cette modernisation est sans incidence sur le dialogue environnemental local, d'une part les décisions soumises à l'évaluation environnementale, c'est-à-dire la quasi-totalité d'entre elles seront bien toujours soumise à consultation d'autre part, toutes les autres décisions feront l'objet d'une information de ce comité de suivi, enfin, je rappelle que la Commission a prévu que ce comité suivi soient également informés de toute évolution dans l'organisation de la concession dans le cadre de la loi climat résilience de 2021 naturellement cette information précieuse, compte tenu du contentieux européen qui a fait que nos concessions depuis bientôt plus de 10 ans est inchangé c'est donc une demande de retrait sinon un avis défavorable. Votre amendement vise à supprimer l'article introduit en commission qui réduit la compétence des comités de suivi de l'exécution des concessions hydroélectriques au seule décision soumise à évaluation environnementale, sur ces bancs la question des concessions hydroélectriques, elle va devoir aborder la question des conflits d'usage et donc on ne peut pas se limiter aux seuls enjeux environnementaux, il nous semble ce comité a un rôle important pour, il a pour objet de faciliter l'information des collectivités locales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et il doit aussi pouvoir aborder la question des différents usages de l'eau ou sur les enjeux de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, donc pour toutes ces raisons, c'est un avis favorable sur ces deux amendements. Donc sur ces deux amendements avec un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement, nous avons une demande de scrutin public du groupe, les républicains. Il va être procédé à ce scrutin public dans les conditions réglementaires. Ah, l'ONU. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, donc le scrutin est clos. Et voici. Le résultat, 343 votants et 343 exprimés

qui le présente. Oui, monsieur le président, c'est là aussi coordination rédactionnelle. Commission. Même chose, je vous propose d'adopter mon amendement de coordination rédactionnelle. Gouvernement favorable pour le 1er sagesse pour l'autre. D'accord. Donc pour l'amendement 567 double avis favorable qui est pour.

la loi énergie-climat a permis la possibilité d'augmenter la puissance des des concessions existantes cependant depuis 2019 malgré le dépôt de dossier par les concessionnaires, aucune de ces augmentations de puissance n'a pu être mis en service pour des raisons procédurales or certaines de ces augmentations de puissance pourrait être mises en oeuvre sans délai, en particulier celle qui ne nécessite pas de travaux pour les dossiers de ce type déjà déposé cet amendement propose donc une autorisation temporaire en cas de situation de tension forte sur le système électrique sans attendre l'aboutissement de la décision pérenne qui pourraient être délivrée elle ultérieurement. Sur cet amendement 21 nos collègues, monsieur le rapporteur. Si Monsieur le Président, la commission a introduit la facilitation de l'augmentation de puissance des des installations hydrauliques concédé qu'elle avait d'ailleurs assoupli en 2019 dans la loi énergie-climat et en 2021 dans la loi climat résilience, elle est donc tout à fait favorable à ce type de dispositif en revanche les modifications proposées par l'amendement ne sont pas souhaitables : d'une part, si la Commission a fait référence à une menace grave pesant sur la sécurité d'approvisionnement, c'est pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 12 août dernier que j'ai déjà évoqué dans laquelle le conseil qu'aussi chez elle, a précisé que certaines mesures nécessaires à la sécurité d'approvisionnement énergétique ne pouvait être compatible avec la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle qu'un cas de menace grave, il est donc pas opportun de remplacer les termes de menace grave par ceux de fortes tensions qui fragiliserait le dispositif d'autre part, l'amendement introduira une référence erronée aux installations hydrauliques qui ne sont pas visés par l'Arctique elle tirer 1 du code de l'énergie, mais de l'article L. 500 tirer 5 nous ne saurions donc plus à quelle installation s'appliquerait le dispositif, c'est donc une demande de retrait sinon un avis défavorable. Madame le Ministre pardon c'était celui celui-là sur lequel j'avais un avis de sagesse. Monsieur Vial, demande de retrait. La réponse est oui. Donc il est retiré, merci Monsieur Gay a déjà défendu son amendement tout à l'heure juste. Monsieur le président, c'est un amendement maintenant de coordination, parce qu'on a voté, on a voté le 400 mètres donc, comme il est, il est identique au 421 j'imagine que j'aurais un avis favorable de Madame la Ministre. Comme je l'ai déjà évoqué le suivi environnemental proposé par l'amendement n'est pas nécessaire tout d'abord, les augmentations de puissance sont déjà de plus d'un tel, suivie de la part du concessionnaire comme de l'autorité administrative de plus le le dispositif proposé prévoit que les mesures soient proportionnées nécessaire limitée et fasse l'objet d'une information des comités régionaux de l'énergie, je demande donc son retrait sinon un avis défavorable. La Ministre, s'il vous plaît. Et alors, non, en fait, là c'est défavorable, parce que c'est pas le même amendement mais vous le savez comme moi, il s'agit effectivement le suivi existe déjà et donc c'est une demande de retrait car satisfait. Je mets au voir retirer. Merci, nous pouvons donc voter sur le seize Sepp Thiès dans son intégralité, qui est pour l'article 16 septs

Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement a pour but, tout simplement de s'enrichir dans nos territoires et en utilisant l'eau sans aucun traumatisme d'une capacité de puissance nouvelle avec les hydroliennes et ce qui est proposé, c'est effectivement d'expérimenter et en plus on a la chance d'avoir des entreprises françaises, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt Madame la Ministre, sur les éoliennes qui étaient fabriqués dans nos Terres le bilan carbone là il est très bon, puisque nous avons et les entreprises dans nos territoires qui sont en capacité de produire ces hydroliennes c'est d'autant plus intéressant que c'est une et NRJ pilotable complètement pilotable c'est d'autant plus intéressant comme je l'ai évoqué qu'il y a aucun traumatisme dans l'eau, pas besoin de faire des travaux, pas besoin d'avoir une canalisation cette hydrolienne est simplement posée sur l'eau et produits cette énergie renouvelable. La ville de commission sur cet amendement, monsieur le monsieur le rapporteur. Monsieur le président, les les hydroliennes fluviales sont un procédé intéressant pour développer l'hydroélectricité sans dégradation du milieu aquatique, or elles sont très peu pris en compte dans les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, qui, c'est plutôt la petite ou la grande hydroélectricité une expérimentation, telle que proposée a le mérite de faire avancer ce sujet, je précise que la commission, tout comme l'auteur de l'amendement ont eu connaissance de plusieurs projets en cours dans nos territoires, c'est donc un avis de sagesse. Madame la ministre.

Donc je vais consulter le Sénat monsieur Gremillet. Commentaire et et de la position du gouvernement, je remercie notre rapporteur. Parce qu'effectivement, contrairement à ce que vous évoquez, il y a un potentiel énorme dans nos territoires. Quand vous voyez ces hydroliennes je peux d'ailleurs. Je me doutais que. C'est pas gros. Une hydrolienne Madame la Ministre, c'est pas gros et ça peut effectivement être pratiquement sur tous les cours d'eau. Et il y a un autre intérêt. On légifère depuis hier. On a beaucoup parlé de photo-voltaïque de renouvelable : éolien. L'intérêt de ces hydroliennes, c'est qu'il y a un mariage complet et très intéressant. Entre la capacité de produire effectivement de l'énergie renouvelable complètement décarbonés et et en plus matériel fabriqué dans nos territoires sur des périodes sur notamment en hiver, nous ce que les cours d'eau sont largement pourvus. Et d'avoir une complémentarité, on était lorsque effectivement il y a une moindre activité au niveau des cours d'eau avec une capacité de production de de photovoltaïque, moi je suis très surpris, vous voyez, on est sur une urgence, on est sur une volonté d'augmenter les capacités de production dans nos territoires d'électricité de décarboner notre énergie il y a des entreprises françaises qui ose entreprendre et et on serait en train aujourd'hui de considérer qu'elle n'apporte aucune réponse alors qu'elles apportent une réponse à ce qui est attendu de notre société et qu'elles apportent aussi une réponse énergétique dans nos territoires, tous nos territoires. Madame la ministre, un complément. juste pour vous dire, moi j'ai rien contre les hydroliennes fluviales mais je, je, je, j'examine et je regarde ce qui ce qui remonte, vous savez que on a aidé un projet de la CNR avec 20 millions va machine qui faisait à peine 2 mégawatts, un niveau de subventions très élevées du pays et ils ont renoncé car ça ne marchait pas, alors peut-être ici sont mal pris un jeu, mais enfin c'est pas de n'importe qui, la CNR et donc je je vois là, on a eu plusieurs tentatives de projets, on a accompagné, on a fait l'expérimentation pour le moment, ça a pas marché maintenant si vous avez des projets sur le territoire qui fonctionne, moi je serais ravi qu'on les rassemble, qu'on les recense et qu'on les retravaille mais pour le moment, c'est pas ce qui est ressorti des différentes expérimentations qu'on a plus ont pu lancer sur ce sujet-là et accompagné par le PIA étant comptable de l'argent public, j'essaie de prendre ce qui fonctionne le mieux dans la boîte à outils qui est à notre disposition. C'est tous ces trucs-là. Je soumets l'amendement au vote avec madame la présidente, avant qu'on vote. Oui, c'est l'heure d'être un peu taquine, mais moi j'ai compris tout à l'heure dans le secteur de l'éolien, qu'il fallait créer le marché par la loi. Pour développer les entreprises, donc je vais soutenir l'amendement monsieur Gremillet et je vais qu'on va essayer ensemble de créer le marché de permettre le marché avec la loi et de trouver les les intervenants après mais je suis un peu taquine à cette heure-ci. Très bien, donc nous, nous nous prononçons sur l'amendement 313 Madame Lienemann, demande la parole auparavant. Oui, moi, je soutiens l'amendement de Monsieur Gremillet parce qu'on a tellement d'exemples où les technologies françaises au début, marche pas forcément très bien, alors on dit : ça marche pas, surtout quand ça vient pas d'opérateur bien bien inséré dans le tissu économique national que du c'est des PME, des groupes comme ça que ça s'est jamais une bonne idée, on fait une expérience puis on dit ça marche pas. Moi je pense que là il y a pas de certitude que ça va bien marcher, mais franchement, ça va pas ruiner la nation de d'élargir un certain nombre d'expérimentations et d'en tirer après coup le bilan, surtout s'il a pas de risques environnementaux et comme le dit Sophie, au bout d'un moment, si vous n'avez pas un minimum de choses qui se déroule et ben, ça ne se développe pas, moi, je crois qu'il faut être, ça va prendre des risques, je me rappelle, on a rencontré le le représentant Monsieur Borrel de d'investissement industriels nous dit faut savoir prendre des risques dans ce pays, ben là il me semble qu'on prendrait des risques mesurés pour une cause qui paraît quand même intéressante donc je trouve que cet amendement mérite d'être soutenu. Merci monsieur le président je soutiendrai également c'est cet amendement, je pense que c'est aussi la problématique des hydroliennes en mer il y a eu des expérimentations qui ne sont pas non plus couronnée de succès, parce que c'est une technologie qui est qui est difficile à mettre en oeuvre, qui est soumise à à à rude à rude épreuve, parce que dans dans le fond de la mer, hé bien là c'est un petit peu différent, on a, on a des galets, on a tout un tas de choses très co très abrasive et corrosive mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner je pense qu'il y a des potentiels et il faut exploiter, il faut expérimenter pour essayer d'arriver hé bien à des résultats plus tangible, peut-être qu'on sera obligé d'abandonner sur certaines choses, mais si on arrête trop vite et bien, on n'aura pas été jusqu'au bout de l'expérimentation. un moment donné, femme appeler un chat un chat, pourquoi toutes ces petites hydroliennes flottantes ou sur les fonds de rivière il y en a quasiment plus en France parce que les seules Start-Up qui à un moment donné, ont été aidées, subventionnées par les états successifs n'ont pas trouvé de débouché, pourquoi, parce que les services de l'État bloque les projets individuels, donc quand il y a pas de marché possible ceux qui ont imaginé des systèmes qui fonctionnent bien, n'a pas pu vendre leurs machines à aujourd'hui la seule hydrolienne flottante qui peut être installé sur le titre hier, c'est une hydrolienne canadienne la plus donc tout ce qui a pu être fait en France, hé ben aujourd'hui ils sont au fond des tiroirs parce qu'il y a pas de débouchés. Je vais mettre aux voix l'amendement 313 avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Bon, qui est contre, il y en a moins, donc, cet amendement est adopté, allez, encore un pour la route.

Si Monsieur le Président, je vous propose adopter mon amendement de précision à. Rédactionnelle la la ministre rédaction. Bien, donc favorable de la commission, ça laisse du gouvernement qui est pour.

Oui, monsieur le président je vais être très bref parce que c'est en droite ligne de ce qui a été présenté, madame la ministre, monsieur le rapporteur et chers collègues, je voudrais vous remercier sincèrement de de cette acceptation d'expérimenter parce que ce qui est proposé, c'est effectivement d'en faire un bilan, et est ce que nous avons envie que c'est c'est que ça marche et pour l'avoir vécu donc tout simplement sur le terrain, je peux vous assurer, Madame la Ministre, que vous serez surprise et que ça apportera un certain nombre de réponses sur nos territoires, donc s'dans même prolongement de la l'activité énergétique à partir des hydroliennes fluviales. La commission monsieur rapporteur. La commission a adopté le principe d'un rapport d'évaluation de l'article 89 de la loi climat résilience qui a apporté dissolution de simplification en matière d'hydroélectricité la ainsi montrer son attachement à l'application des lois, celle-ci progresse puisque le décret relatif au médiateur national de l'hydroélectricité et au portail national de l'hydroélectricité ont bien été pris en juillet dernier l'amendement proposé vise à intégrer les hydro-le yen fluvial sujet nouveau mal appréhendé par le droit au Champ de ce rapport d'évaluation, c'est donc un avis de sagesse. Madame la ministre, l'avis du Gouvernement défavorable, défavorable, monsieur Gilles demandé à s'exprimer. Ce sera très rapide, mais je suis très surpris, monsieur le rapporteur, puisque, pour le coup, vous acceptez un rapport parce que depuis, depuis des heures à chaque fois que vous intervenez, vous nous dites que le Sénat, par principe, n'accepte pas de rapport et alors là, vous acceptez un rapport donc je considère que le principe du Sénat est tombé et que donc on pourra que c'était des rapports. ça ouvre les vannes, madame la présidente. Merci Monsieur le Président, alors monsieur Julien, je vais vous rassemble, je vais vous rassurer, on ne va pas faire tomber le principe voilà et je vais demander à mon collègue Daniel Gremillet peut être malgré l'avis de sagesse de la commission et je vais lui demander à mon titre à titre personnel de peut être retiré son amendement et lui proposer que cette évaluation, nous la fassions dans le cadre des travaux de la commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Madame la présidente. Cette proposition me va très bien. C'est même mieux. Compte tenu que la avant monde précédents, a été voté, ce qui était important, c'était de lancer une expérimentation, ce qui était important, c'était de pouvoir en tirer le bilan, sur 3 ans, ce qui était important, c'était de pouvoir le développer sur les territoires et effectivement la richesse et le travail de la commission économique Madame la Ministre vous prouvera l'intérêt d'avoir osé aujourd'hui d'entreprendre et de donner confiance à des entreprises qui investissent et des entrepreneurs qui investissent dans nos territoires avec de l'hydroliennes fluviales. Dans la cloche qui vient : il a retiré ne nous empêche pas de nous prononcer sur la sur l'article 16 oct Yes nouveau, ce sera le dernier vote de cette fin d'après-midi, qui est pour l'article. Contre. Il est donc adopté je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, qui comporte maintenant cent Donc bon courage il a séance est suspendue.